L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement numéro 74 rectifié au sein de l'article 9. Donc pour l'article 74 rectifié la parole à Madame Préville. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je propose d'ajouter à cet article 9 un alinéa précisant les friches qui peuvent être concernés, parce que les friches sont bien différentes, alors que, il y a un aspect très négatif au mot friche. Et lorsque l'arrêt de l'exploitation économique ou militaire est très ancien, le concept de friches pourraient être revus parce que il serait nécessaire de prendre en compte la biodiversité qui est souvent présente sur ces zones qui ont été trop dit trop rapidement qualifié de friches. Et correspond souvent à un plan écologique, il y a des zones de libre-évolution comme j'en ai déjà parlé précédemment hier et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques et là je ne parle pas de renaturation mais de tenir compte de l'état des lieux de ces terrains, à savoir que la nature, il a repris ses droits et que de fait, elles sont un réservoir de biodiversité dans cet amendement, je vise également à imposer la réalisation d'un inventaire national de CDS de ces friches, sur la base de données actualisées par ailleurs j'inclus également le fait que le dispositif relatif au site naturel de compensation qui a été introduit par l'article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la bière biodiversité de la nature et des paysages, a vocation à compléter le panel d'outils à disposition des maîtres d'ouvrage pour remplir leur obligation de compensation donc j'exclus de fait, ces sites de compensation et vise notamment à répondre aux difficultés de mise en oeuvre effective de la compensation liée à la disponibilité, il semble essentiel que ces sites identifiés comme site naturel de compensation puisse rester disponible pour de telles mesures de compensation présent amendement propose donc de rajouter une exclusion par principe de ces zones merci. Oui, Monsieur le Président, cet amendement est satisfait par le texte proposé parce que, après le passage en commission sont bien les sites dégradés qui pourront faire l'objet d'une dérogation lorsque celui-ci est techniquement réalisable exclusion décide identifié comme site naturel de compensation proposée par cet amendement me semble donc satisfaite: c'est un avis défavorable. Madame la Ministre défavorable. Il y a un double avis défavorable, il n'y a pas de demande de prise de parole, on passe au vote. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 52 rectifié bis monsieur Vial. merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un d'un d'un amendement de cohérence, nous sommes là pour essayer de, de développer l'installation de panneaux photovoltaïques et, comme ça a été permis dans le reste de la loi, il y a un gisement qui, elle, est ce qu'on appelle les délaissés sur les aéroports ou les aérodromes de de terrain qui ne peuvent être ni agricole ni naturel, qui ne peuvent pas avoir d'autres, d'autres usages et qui permettrait de, d'accueillir des installations photovoltaïques hors la loi littoral interdit ce type d'installation et donc mon amendement prévoit par dérogation à la loi littoral, comme cet cet article le le permet, nous puissions autoriser les les oraux, les aéroports situés en zone littorale pour utiliser ces délaissé et mettre en place des panneaux photovoltaïques, ils ont organisé une une étude qui a été fait en en 2013 par l'aviation civile qui qui détermine justement le le potentiel de ces zones dans les aéroports, l'ensemble des aéroports de France auront accès à ce ce mode de développement, on a un certain nombre d'aéroports, tout le monde pense à celui de Nice, du Havre, mais aussi à celui du Bourget du Lac au au bord d'un d'un lac naturel qui est classé en loi montagne et loi littoral l'objectif de cet amendement est me semble-t-il cohérent de permettre à ses aéroports comme aux autres, de pouvoir mettre en place des panneaux photovoltaïques, sans que ça, ça porte atteinte à l'esprit de la loi littoral. Monsieur le rapporteur. Oui, jusqu'à présent, cher collègue, votre amendement évidemment je, je, j'ai souscrit et je le partage, il est déjà satisfait parce que nous avons intégré dans le système de dérogation à la loi littoral à l'article 9 puisque ces sites sont considérés comme des sites dégradés, ils n'ont pas d'autres destinations et et pourront donc être couvert l'amendement est donc satisfait. Madame la Ministre. Même avis : demande de retrait ou avis défavorable.

Il y a un amendement retiré donc 2 amendements en discussion commune le 1er présenté par Monsieur Gremillet. Le 497. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement propose tout simplement d'avoir un avis conforme de la Cdpenaf concernant la station photovoltaïque. Monsieur Dantec, le deuxième. Oui merci monsieur le président, c'est un amendement qui va dans le même sens, mais l'axe avec Daniel Gremillet connu mais moi je ai pas j'ai pas rajouter agricole friche tout court, je ne vois pas pourquoi on aurait pas un avis conforme sur les deux donc j'ai bien noté hier que le Sénat avec des majorités très larges mettent des avis conforme, donc là je crois qu'on est dans la même logique, donc, on rajoute un avis conforme, ce qui correspond aussi au fait que si vous vous rappelez, hier, hein, on, on, on est arrivé à la conclusion que ça n'était pas dans l'émission du Conservatoire du du littoral,

un avis de la commission sur le rapporteur. Oui, c'est cet amendement sa maman évoque des parcelles agricoles et pastorales, alors que l'article 9 portent sur des sites dégradés, par ailleurs que l'adoption de cet amendement conduirait à supprimer la ville là c'est NPS sur la décision d'autorisation pour les installations qui ne serait pas implantés sur des parcelles susceptibles d'une mise en valeur agricole au pastorale, c'est-à-dire pour l'essentiel des cas prévus par l'article 9, c'est donc un avis défavorable, et puis pour celui de de notre collègue Ronan Dantec, quand on a examiné cette disposition dans la loi climat et résilience et dans le cas de la proposition de loi que j'avais porté, nous n'avons jamais prévu d'avis conforme de ces BMPS, je ne souhaite pas revenir sur cet équilibre, donc un avis défavorable. Madame la Ministre avis défavorable sur les deux amendements. Donc un double avis défavorable sur les deux amendements monsieur Gremetz. Monsieur le président, je leur tire. OK Monsieur Dantec, oui, je vais le retirer. il est retiré, donc les deux amendements sont retirés, ensuite nous avons 3 autres amendements en discussion commune 3 amendements identiques. Le 1er monsieur le présent amendement vise à garantir que lorsqu'ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à le littoral, les projets d'installations photovoltaïques sont réversibles et fassent l'objet de garanties permettant leur démantèlement, dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des soldes, les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respecté et l'installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols, il a fait reculer le foncier agricole. Merci l'amendement suivant identique, madame Saint-Pé. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, l'amendement vient déjà être exprimé, donc il est déjà défendu merci président. Merci monsieur Gremillet pour le 3ème défendu avis du rapporteur. sur le site agricole le reste de la réglementation et la législation s'applique. Madame la Ministre même avis. Donc un double avis défavorable, les amendements sont maintenus ou. Retiré. Tirer. Président je j'ai pas allonger le débat, je vais le retirer mais c'est un vrai sujet quand même le fait qu'il est l'engagement à la certitude que celui qui implante déconstruisent en totalité, on aura le sujet plus tard encore dans le débat sur ce texte, donc j'ai bien entendu ce qu'a dit notre rapporteur, je leur tire, mais c'est un sujet, il est pas si simple que cela, et il donne quand même quelques sécurité sur nos territoires. Merci, cher collègue, donc les amendements sont retirés le 223 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement de coordination mais je me dis : pas de l'issue fatale de cet amendement, en effet, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable à remplacer la notion de friches par celle des sites dégradés pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie solaire, hydrogène renouvelable ou bas-carbone couplé avec ses ouvrages ainsi que d'installations de stockage d'énergie en dérogeant à la loi littoral, telle est l'objet du présent amendement qui conforte l'extension adopté en commission, cela permettra notamment d'inclure les terrains éligible aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, soit 100 francs 12 projets de centrales solaires sur des terrains dégradés actuellement. Avis du rapporteur, un avis favorable à cet amendement de coordination. Madame la ministre, non, c'est un avis défavorable la notion de sites dégradés et je l'ai déjà dit dans des amendements précédents, c'est une notion potentiellement très large, qui n'est pas défini par le code de l'urbanisme à la différence de la notion de friches qui figure à l'article L. 111 26 et comme je l'ai défendu hier a potentiellement cette notion fragilise cette dérogation à la loi littoral dont vous savez qu'elle est extraordinairement scrutés par le Conseil constitutionnel. Monsieur Dantec. Donc un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président, moi je vais dans le sens de madame un un ministre

potentiellement un un risque en termes juridiques, mais derrière il y a une autre question qui fait écho au débat qu'on a eu hier soir vous en rappelez tous autour de la Valduc et des étangs Camargue et tous les sites dégradés n'ont pas vocation à accepter d'autres activités humaines un certain nombre de sites dégradés ont vocation à être repris pour la biodiversité et je pense que la la notion de sites dégradés est assez dangereuse, surtout qu'on est quand même sur la la loi littoral, et je pense que le terme friche effectivement correspondait mieux et donc on ne peut pas voter évidemment l'amendement ni l'article. Bien monsieur Corbizet. C'est un moment, on ne m'appartient pas, donc je l'ai défendu il y a pas, du moment où la commission l'a examiné la valider, je remercie le rapporteur je maintiens cet amendement.

Dans les mains, s'était levé tardivement mais j'avais vu que le groupe Les Républicains et voter voté contre, donc qui qui qui est Qui s'abstient, donc il est adopté, nous passons au vote sur l'article 9 qui est pour l'article 9. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté, donc des amendements après l'article 9 5 amendements identiques le le 1er présentée par Madame Préville. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement propose d'étendre la dérogation au principe de continuité dont bénéficient les stations d'épuration des eaux usées aux travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations afin de favoriser l'autonomie énergétique de ces sites. en vue de leur permettre l'autonomie énergétique, je vous remercie.

monsieur renonce Arazi défendu monsieur le rapporteur. Monsieur le président je vais prendre quelques instants pour répondre, évidemment, pour ces cinq amendements, il me semble qu'ainsi rédigés ces amendements viendrait à déroger au principe d'urbanisation continuité des villes et villages existants zone littorale pour toutes les installations de panneaux photo-voltaïque, ce n'est évidemment pas l'intention de l'article 9 qui a prévu des encadrements de permettant d'autoriser sa session que sur les sites dégradés, l'objet de discussion précédente, il me semble que l'intention qui vient d'être affirmée des auteurs, c'était plutôt d'autoriser des panneaux sur les stations d'épuration des des eaux usées situé en zone littorale me semble donc que ces amendements sont satisfaits dans leur intention par l'article 9, telle que modifiée par la commission qui permet des dérogations au principe d'urbanisation continuité des villes et villages existants pour l'installation de panneaux solaires sur les sites dégradés, en effet, si les stations d'épuration sont considérés comme des sites dégradés, les installations solaires pour naturellement il être autorisé au titre d'article, là, c'est donc un avis défavorable. Madame la Ministre même avis. Donc même avis un double avis défavorable, donc je l'ai sous, mais on voit qui est pour.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à faciliter dans les territoires ruraux déjà urbanisée au sens des PLU et des Scott notamment les bâtiments industriels les l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une auto-consommation, or l'installation de tels dispositifs est aujourd'hui considérée comme une extension d'urbanisation aussi par cet amendement, je vous propose une dérogation au principe de continuité d'urbanisation dans les cas de dispositifs de production d'énergie sur le terrain d'assiette de l'entreprise visant sa consommation directe, je vous remercie. merci monsieur le président de la Ministre donc le caractère stratégique que revêt le développement de la production d'énergie renouvelables impose de saisir aujourd'hui toutes les opportunités, à ce titre, les secteurs déjà urbanisés, autre que les agglomérations et les villages, identifié par le schéma de cohérence territoriale et délimité par le plan local d'urbanisme, on devrait pouvoir être mobilisés également, or actuellement sur nombre de communes littorales existe des équipements industriels publics ou privés en zone d'organisation diffuse plusieurs de ses installations sont très consommatrices en énergie des demandes de se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d'assurer une forme d'autonomie énergétique de l'équipement, ces panneaux étant considérée comme une extension de l'urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusé, quand bien même les dispositifs planterai sur Parking ou autres zones artificialisées directement adjacentes au site afin de promouvoir au plus vite l'indépendance énergétique sans aucun impact sur les Terres agricoles ou naturels, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d'urbanisation dans le cas de dispositifs de production d'énergie sur le terrain d'assiette de l'entreprise visant à sa consommation directe. Avis de la commission sur ces quatre amendements identiques. Monsieur le président, une opération de de consommation sur le terrain d'assiette du producteur nécessite-t-elle une dérogation au principe d'urbanisation continuité des villes et villages existants, comme le proposent ces amendements, j'ai mis un point d'interrogation, j'en doute, puisque les installations nécessaires à l'eau de consommation sont souvent installés directement sur les habitations continuité ou des bâtiments ont continuité directe de celle-ci, donc je m'en remets à l'avis du gouvernement, parce que, a priori sur ces espaces sur ces assiettes là il devrait pas y avoir de c'est Madame la Ministre. Et effectivement, je rejoins le question non, en tout cas l'analyse de monsieur le rapporteur, a priori, ce n'est pas une disposition qui va ouvrir beaucoup d'espace, puisque l'autoconsommation en règle générale, se fait sur toiture ou à proximité d'habitations, et en l'occurrence, votre amendement va élargir à nouveau les dérogations à la loi littoral pour les installe la loi littoral, et vous savez que nous estimons qu'il faut encadrer ces dérogations, compte tenu des enjeux de la charte de l'environnement et du risque d'inconstitutionnalité des dérogations que nous prenons. Donc un avis défavorable du gouvernement, monsieur le rapporteur. Le coup. Donc double avis défavorable je soumets les amendements voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés. L'amendement 355 Madame DeMarco Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, les défrichements forestier, dit à l'installation de centrales photovoltaïques sont de plus en plus nombreux, notamment dans le massif landais ou plusieurs milliers d'hectares sont concernés, par exemple, la Soka Gironde des énergies Titi siens souhaite construire la plus grande centrale de solaire d'Europe sur plus de 1000 hectares de pins après les violents incendies de cet été, de nombreux propriétaires forestiers sont également démarchés par des sociétés qui cherche, installer des fermes photovoltaïques sur les parcelles brûlées, la forêt est également un réservoir de biodiversité permet d'absorber du CO2 atmosphérique, il est donc nécessaire d'évaluer les conséquences environnementales de ses installations, sans oublier que la filière bois est une ressource essentielle pour nos territoires avec plus de 50000 emplois rien qu'un Nouvelle Aquitaine alors que de nombreuses questions restent sans réponse, nous devons rester vigilants, le rapport qu'une demandons permettra d'éclairer la situation et de légiférer en connaissance de cause. Merci, cher collègue à vie de monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, chers collègues par par principe, nous sommes plutôt défavorable, rapport, même si le sujet de celui-ci nous intéresse en en plus haut lieu puisque nous avons à la fois avec la commission d'affaires et notre commission mis en place une mission d'information sur sur ce cette thématique et cela devrait déboucher sur une proposition de loi qui arrive en novembre qui sera déposé par notre collègue ici présent Jean Madame Loisy monsieur Martin Monsieur Reitmans dans le courant du mois, donc n'anticipons pas les la proposition soit de loi se s'étudier et puis nous nous intégrons ces questions là, donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. c'est également un avis défavorable je rappelle que les dispositifs de soutien mis en place aux projets photovoltaïques, par le gouvernement, interdisent déjà les projets implantés sur des sites ayant nécessité un défrichement donc ça je pense que c'est important de le rappeler, par ailleurs, il me semble que votre questionnement tourne autour de l'utilisation de sites qui aurait été déchets Frichet, ça peut être pour des panneaux photovoltaïques, ça peut être pour autre chose, il me semble, il faut prendre le sujet sous cet angle est pas stigmatiser l'implantation de panneaux photos vol. A fortiori, s'agissant d'une d'un usage qui est démontable et qui par ailleurs contribue à lutter contre le dérèglement climatique et vous le savez, un observatoire des énergies renouvelables en forêt sera lancée par l'ONF dans les prochaines semaines, donc il me semble que votre amendement est satisfait. Donc 2 avis défavorables je soumets l'amendement voit qui est pour. Pardon il est retiré, pardon, excusez-moi. Bien on continue donc en attaquant les amendements de l'article 10 donc, le 533 monsieur Houlgate. Merci monsieur le président, la loi montagne protège les espaces afin de limiter le mitage et l'étalement urbain acte ainsi le principe de l'urbanisation en continuité du bâti existant ce principe prévoit néanmoins des exceptions qui sont mesurés, notamment pour les communes qui sont couverts par un Scott ou un PLU, dans le cadre d'une étude de discontinuité, l'objectif est bien de garantir un équilibre entre protection et aménagement des espaces de montagne, or le projet de loi prévoit que la carte communale, les communes non couvertes par un Scott pourra comporter une étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque en discontinuité cette mesure ou plaît à l'absence de planification territorialisée, risque de conduire à un développement désordonné des implantations, tout en aggravant le mitage des territoires de montagne par ailleurs Setanta risque de ne pas aller dans le sens d'une meilleure appropriation des projets solaires par les habitants aussi notre amendement propose de limiter la portée de l'article 10 aux installations qui constitue un équipement collectif et de privilégier dans les partis non-urbanisées, des communes, la pose de panneaux solaires sur le bâti existant. avis de la commission. à avoir une PPL sur l'agrivoltaïsme et intégrer cette question là, puisque on a vu le déploiement d'un certain nombre d'installations justement sous couvert d'équipements collectifs dans les dans les règles d'urbanisme, donc c'est un avis défavorable à à cet amendement.

c'est un avis défavorable car cet amendement est déjà satisfait par le droit commun de l'urbanisme et avis favorable sur l'amendement de coordination de monsieur le rapporteur. Alors donc, l'amendement est retiré et ensuite, nous avons un amendement de la de la commission qui est un amendement de coordination que vient d'évoquer monsieur le rapporteur, et auquel le gouvernement donne un avis favorable ou qui est pour cet amendement. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, donc nous passons au vote sur l'article 10 qui est pour l'article 10.

plus tôt dans le département que vous connaissez bien ah projet primé par votre ministère une centrale solaire de 32000 panneaux photovoltaïques, sur 30 hectares a été inauguré en particulier installé sur une ancienne friche d'enfouissement de déchets ménagers, mais que de temps perdu par rapport aux règles du PLU, voilà pourquoi ce présent amendement propose de permettre de déroger aux règles. Des PLU relatives à l'emprise au sol à la hauteur à la plantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'implantation de centrale centrale photovoltaïque au sol sur des terrains relevant d'une activité de gestion de déchets non dangereux, et cetera présente peu d'enjeu en terme d'articulation des sols, ce qui constitue un foncier mobilisable pour accueillir des projets photovoltaïques, donc, nous avons trois amendements en discussion commune le suivant monsieur Chevreau. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les installations de stockage de déchets non dangereux sont conçus pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des quasi-aménagés dans des conditions de sécurité optimisée optimisée pour pour l'environnement, donc les quasi en post-exploitation constituent des des surfaces disponibles qui pourraient être utilisés dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment pour la préservation de la qualité des des sols donc ces sites pourraient être équipé de panneaux photovoltaïques, les acteurs de la gestion des déchets, estime qu'il y a un potentiel de 300 gigawatts à l'horizon 2030 et 600 gigawatts à l'horizon 2040, donc c'est un potentiel important et à l'heure où il faut agir pour notre climat et développer la production énergétique cet amendement propose de lever les freins qui existent aujourd'hui au déploiement de ces panneaux Photoways voltaïque dans les anciennes zones de centrales de Centre de stock de stockage de déchets non dangereux, je vous remercie. Merci, et le troisième, le 380. Madame avait il est défendu. Il y a un monsieur le rapporteur, avis sur ces trois amendements. ne me semble pas empêché dans l'absolu, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites de stockage de déchets dangereux, en tout état de cause si les PLU limite ponctuellement ou limité aujourd'hui ponctuellement l'installation de panneaux voltaïque sur saisie une modification du PLU par la procédure simplifiée ouverte par l'article 3 de ce projet de loi que nous avons voté hier sera possible et constituera donc une réponse satisfaisante à la problématique soulevée par ces différents amendements, c'est donc un un, une demande de retrait sinon un avis défavorable. Madame la Ministre. C'est un avis de sagesse parce que je pense que l'exemple donné par monsieur le sénateur, Corbizet montre bien qu'il y a des frottements et donc. C'est vrai que l'analyse juridique apportée par monsieur le rapporteur, paraît de bon sens, mais néanmoins on voit que sur le terrain, ça bloque, et donc je pense que ça mérite d'être regardé de plus près. Donc, avis de sagesse du gouvernement, nous allons procéder au vote, donc les amendements seront maintenus, d'abord. Oui, ils sont maintenus. Donc l'amendement de Monsieur Qui est favorable. Qui est contre.

les deux autres tombes non puisque le 1er est adopté. Donc après

il introduit un nouvel article au sein du code de la santé publique, qui a dit que les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l'article L-1321 2 dans la zone de protection rapprochée que si des t'apporter la preuve d'un risque d'une particulière gravité pour la qualité des eaux, cela permet de renverser le mécanisme en faisant de l'autorisation, le principe de l'interdiction l'exception en la plaçant sous des conditions strictes que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier par ailleurs il est prévu que les préfets mon différents, les déclarations d'utilité publique, assistante par une procédure simplifiée, dans un délai d'un an. vis du rapporteur. Soir. Cet amendement qui permettrait le déploiement d'installation voltaïque photovoltaïque à proximité des zones de captage sauf si ai apporté la preuve d'un risque d'une particulière gravité pour l'accueil des eaux ne me semble pas conforme au principe de précaution, ils pourraient en effet y avoir des risques induits par l'implantation d'installations photovoltaïques à proximité des zones de captage je pas certain qu'il faille prendre ces risques pour un bénéfice très limités en matière de foncier libéré travaillant sur toutes les surfaces disponibles sur les toits sur les espaces qu'on a largement évoqué, avant d'aller sur ces zones un peu plus sensible en terme de captage, c'était donc un avis défavorable. Madame la Ministre, c'est également un avis défavorable. merci, donc un double avis défavorable, l'amendement est maintenu, il est retiré, nous passons donc à la discussion de l'article onze avec trente-six amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Donc le premier le onze rectifié monsieur saumon. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement prévoit une alternative au dispositif des ombres hier par un revêtement de surface qui intègre un procédé de production d'énergie renouvelable sur la totalité de leur surface en effet cette technologie permettent de assurer l'éclairage public, le chauffage, le refroidissement de bâtiments à proximité, ainsi que le refroidissement de l'air ambiant et j'ai un témoignage particulier parce que, dans la Somme, on a fait ça dans un cours de collège. Alors ensuite donc, 2 amendements identiques le 54 rectifié Monsieur Vial. La coalition. Oui merci monsieur le président, madame la miss, je suis content que cet amendement arrive au début de la discussion parce que ça va nous permettre probablement d'avoir un éclairage sur ce ce dont on va vraiment débattre mon amendement parle des parcs de stationnement, tels qu'ils sont rédigés dans dans l'article et propose de rappeler de de remplacer la notion de parcs de stationnement extérieur par surface extérieure dédiée au au stationnement, pourquoi, parce que le la notion de parcs de stationnement renvoie au code de la voirie routière et et donc au stationnement payant, tandis que la notion d'aires de stationnement renvoie des surfaces de stationnement qui peuvent être gratuite alors que parcs aires de stationnement dans le sujet, c'était, c'est par exemple une compétence que peuvent avoir les métropoles où les agglomérations et ne fait pas de distinction de différentes une parc un parquet un aire de stationnement

un parc de stationnement gratuit, c'est-à-dire un Parking de supermarché ne serait pas soumis à à ce ce type d'obligations quant à un Parking payant qui appartient à un bailleur dans une résidence de tourisme ou sur sur ou sur un site touristique protégé qui serait payant lui il serait il

le l'amendement suivant c'est madame Saint-Pé. Oui président amendement dit défendue par l'orateur précédent merci. Merci, ensuite le 82 rectifié monsieur Cabanel. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le présent amendement propose de préciser les obligations instaurée à l'article onze visant à équiper d'envoyer un photovoltaïque, elle les partir les parkings extérieurs, nous proposons de remplacer la notion de parking extérieur partielle de Parking de surface et de cibler l'obligation sur les véhicules légers, afin de prévenir tout problème d'interprétation, il est en effet souhaitable d'exclure les parcs de stationnement dit aérien

Oui, il s'agit de compléter la définition de parcs extérieur pour bien avoir une une unité, d'un seul tenant, parce qu'on pourrait très bien imaginer des parkings, on atteindrait la surface mais avec un émiettement sur plusieurs zones, et à ce moment-là on surenchérit serait le coût des investissements.

pour nous de définir des parcs a su faire des parcs de stationnement accueillant les ombrière photovoltaïque. Plutôt en mètre carré quand nombre de places, alors j'entends bien les autres amendements qui ont été produits, mais ça nous paraît plus rationnel, plus compréhensible de le définir mètre carré et par conséquent en républicain que nous sommes notre préférence va au système métrique merci. Oui, merci Monsieur le président, tout en étant très sensible à l'intervention précédente, je pense que mètres carré ça aurait peut-être plus lisible, mais pour l'instant dans le texte, c'est un nombre de places, donc nous on on propose de réduire ce nombre de places de 80 à 50. Les cinquante quand on considère que, entre la place de parking et la voirie, c'est à peu près vingt mètres carrés cinquante ça tombe à peu près sur 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés pour les surfaces bâties c'est justement là où on met, on impose du photovoltaïque, donc le 50 places serait assez logique parce qu'on par rapport à ce qu'on a déjà pu voter sur des surfaces bâties. rectifié, madame Lavarde. Oui, il vise en fait à exclure les aires de stationnement qui sont en fait des airs de logistique, sur lesquels on a des opérations de manutention lourde avec notamment des prises en hauteur qui sont incompatibles avec l'installation de d'ombre Ensuite, le 119 rectifié, je ne sais pas qui veulent défendre personne visiblement donc il est défendu. Ensuite, le 180 rectifié madame Sempé. Oui, monsieur le président, cet amendement vise à exclure explicitement les aires où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement industriel et logistique du Champ de l'application de l'article Merci ensuite 2 autres amendements madame Lavarde le 95 rectifié. Oui, là il s'agit d'un amendement qui vise en fait à rationaliser le coût des investissements puisqu'on a une unité foncière sur laquelle on peut avoir et des bâtiments et une aire de stationnement, l'aire de stationnement peut être soumise à l'obligation d'installations de production d'énergie renouvelable selon quoi, on est tout à fait d'accord, par contre, il peut être plus pertinent que les installations soient installés sur les bâtiments clos couvert qui sont sur la même unité que sur l'aire de stationnement, donc ça vise en fait à pouvoir autoriser le transfert du lieu d'implantation des investissements de production.

permet d'exclure les parkings essentiellement destinée aux poids lourds de l'obligation nombreux hier en raison des difficultés des difficultés techniques et de sécurité puisque les poids lourds nécessite une surface de manoeuvre très importante.

Oui Mercier président l'installation d'Brière viendrait réduire le nombre de places disponibles lorsque il s'agit d'entreprises qui ont des camion volumineux et donc le nombre de places disponibles seraient réduites d'environ 10 % et limiteraient d'après ce qui est prévu, les capacités des entreprises du transport logistique merci. Merci le 465 rectifié monsieur Corbizet ou monsieur Cabanel. Défendu. Monsieur Dantec pour le 297.

L'amendement proposé rétablit la rédaction initiale du texte, s'agissant des cas d'exonération car le contrôle de ces dérogations se fait par le représentant de l'État dans le département, il supprime la disposition tendant une répartition par la commune des ombrière de leur territoire, car cette disposition est inapplicable dans la mesure où il sera impossible de mutualiser les obligations d'installation d'ombre entre des propriétaires de parking extérieur différents. madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président, cet amendement vise à appeler l'attention sur un certain nombre de parcs de stationnement qui peuvent avoir des utilisations diverses autres que le stationnement sur une partie du temps et donc l'amendement vise à étendre la possibilité d'exception, aucun des parcs de stationnement accueillir par exemple des festivals, des fêtes foraines des cirques qui ne pourrait plus s'y installer, si on a un sale des ombres hier. Merci, ensuite le 246 rectifié monsieur corps OK, défendu le 460 17 rectifié Monsieur Jeunet aussi. Oui, merci Monsieur le Président l'amendement déposé par là même, Borchio Fontimp, vise à peu près la même chose que ce qui était visé, l'amendement précédent, simplement le le l'objet est un peu différent mais il. il. S'agit que les parcs de stationnement des gestionnaires de sites événementiels qui sont soumis à de nombreuses conditions d'exploitation spécifique à leur domaine puissent être pris en compte et donc on en serait en plus de contraintes techniques, les contraintes d'exploitation. Merci, ensuite le 41 rectifié, monsieur Sautarel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à prendre en compte les contraintes des exploitants aéroportuaires dès lors que celles-ci peuvent démontrer que l'obligation prévues au présent article ne pourraient être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables en raison des contraintes liées aux changements d'affectation des parcs de stationnement et l'adaptation du service public aéroportuaires, les exploitants aéroportuaires identifie des surfaces qui pourrait être MUTAP dans un horizon défini pour assurer l'adaptation du service public aéroportuaire et, le cas échéant, répondre aux exigences du cahier des charges des concessions des délégations de service public, cela les conduit notamment envisager des changements d'affectation de certains parkings extérieurs, or le temps de retour sur investissement de l'installation dans Brière intégrant les panneaux photovoltaïques étant long ces ombrière peuvent bloquer de tels développements futurs, au détriment des services publics aéroportuaires, je vous remercie. monsieur le président, même la Münich collègues cet amendement permet aux gestionnaires d'aéroports qui peuvent disposer d'autres surfaces disponibles toiture ou au sol, d'installer des panneaux photovoltaïques dans des conditions économiques plus intéressantes qu'en nombre hier de c'est un amendement qui rejoint celui qui a été présenté par mon collègue.

Monsieur Monsieur le Président, cet amendement vise à à limiter le l'obligation d'installation de saison Brière dans les zones dites naturelles ou environnemental puisque des aires de stationnement, on en trouve évidemment en milieu urbain, mais on en trouve aussi en milieu de montagne en milieu naturel en zone protégée en dans dans des parcs naturels nationaux ou ou à proximité de sites touristiques, il il y a 2 caractéristiques : il y a la capacité de raccordement de de ces zones, puisque c'est, c'est aussi l'intérêt de produire de l'électricité, c'est pouvoir la la la, raccordé au réseau l'utiliser sur place qui n'est, tout ce j'imagine quelques exemples en tête ou ce n'est pas possible et deuxièmement la la la qualité aussi de de Cécile con dénaturerait là aussi on pourrait prendre un certain nombre d'exemples mais je suis sûr que vous les avez tous en tête de sites naturels sur lesquels artificialiser de cette manière le le site poserait de gros problèmes, donc je propose de de rajouter après les exceptions prévues par l'article aux sites patrimoniaux de rajouter patrimoniales et environnementales, ainsi que relatives aux sites naturels et aux paysages. Merci monsieur saumon. Oui, dans la même veine que Cédric c'est de préciser aussi qu'il convient de concilier l'ensemble des objectifs environnementaux et que cette production ne doit pas venir à l'encontre des objectifs d'infiltration des eaux pluviales, là où il y a déjà eu des équipements fait en ce sens.

consacré par la loi climat résilience le le principe de Zahnd vise à adapter les règles d'urbanisme existantes pour lutter plus efficacement contre étalement urbain et donc, pour atteindre cet objectif de nombreuses surfaces dédiées au stationnement n'ont pas vocation à être pérennisés, il faut donc pouvoir les exclure de de ce dispositif en équipant ses parcs dont photovoltaïques sur la totalité de leur surface ainsi que des revêtements de surface, nous favoriserons ainsi donc la la perméabilité l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, donc je vous remercie.

ce sont d'ailleurs des investissements qui obtiennent d'excellents résultats résultats pour lutter contre les îlots de chaleur. Merci monsieur le président, le président Internet demain vise à supprimer la possibilité de panacher les obligations d'installation donc brillant photovoltaïques sur les parkings extérieurs de plus de 80 places introduite à une commission le permet aux collectivités compétentes de répartir les hommes brouillard sur les différents parcs de stationnement situés sur leur territoire pour tenir compte, j'ai des difficultés techniques d'implantation ou des coups d'aménagement, cette mesure peut générer des conflits et introduit de la complexité, y compris pour les collectivités territoriales, alors que le gestionnaire de parkings pourra bénéficier de dérogations pour tenir compte des contraintes techniques de sécurité architecturale, patrimoniale ou économique. Merci, un amendement de la commission le 670 présenté par monsieur Mandelli. de répartir les obligations prévues par l'article 11 entre les parcs de stationnement situés sur leur territoire ne vaut évidemment mais c'est mieux de le préciser que pour les parcs de stationnement dont elles sont gestionnaires ou propriétaires bien sûr. Merci le sens être rectifié madame Truchet. Ce. Si Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui permet de repousser le délai de mise en conformité des parkings à 2030 dans un souci de faisabilité le financière logique tic, pour les entreprises.

existant au 1er juillet 2023, ce délai de 5 ans pour les parkings de moins de 400 places et de 3 ans pour les parkings de plus de 400 places, or avec mon amendement, si vous le votez, j'en suis convaincu, ça permettra de supprimer ces délais qui implique une entrée en vigueur très tardive, soit en 2000 28 et ça nous permettrait donc déjà de produire toute de suite entre 6 7 et et 11 gigawatts merci.

on prolonge un délai, c'est-à-dire qu'on on propose de prolonger de 3 à 5 ans le le délai de possibles pour la réalisation de ces équipements pour les pour les stationnements supérieur à 400 places et de 5 à 7 ans pour, pour, pour les autres, pourquoi, tout simplement parce qu'on veut que ça marche que aujourd'hui mettre en place des équipements de cette taille là sur des des parkings de 500 600 ou 1000 places ça nécessite non seulement des moyens de la trésorerie, ça nécessite qui qui qu'il faut rassembler mais ça nécessite aussi d'avoir des entreprises qui soit en capacité de les installer.

il faut qu'on ait le temps, les acheminer Chine ces panneaux photovoltaïques, Madame la Ministre, donc je, je, je propose que, si on veut effectivement augmenté la la la capacité de production et si on veut donner à cet article un peu de sens, il faut aussi donner des délais qui soit compatible avec les règles d'urbanisme d'appels d'offres, les règles financières mais aussi à la filière industrielle et notamment la nôtre de de pouvoir répondre à ces projets. Merci, et enfin un amendement identique toujours madame. Donc il est défendu merci président Karoutchi, donc nous avons trente-six amendements en discussion commune, je vais demander l'avis de la commission pour commencer. Merci monsieur le président, le nombre d'amendements et leur diversité traduit bien l'intérêt chacun apporté à ce sujet, qui méritait effectivement d'être éclairci. Nous avons souhaité conforter le dispositif de couverture des parkings proposée par le gouvernement, la rédaction proposée dans le texte initial soulevé néanmoins plusieurs difficultés, c'est pourquoi nous avons procédé avec la commission à faire écho il récuse réécriture intégrale de l'article onze pour faciliter l'application du dispositif pour les acteurs, sans toutefois en réduire la portée, cet équilibre co-construit avec la commission faire écho me semble plutôt bon je vais pas dire le contraire, faisons en sorte de ne pas trop le toucher pour l'indépendance énergétique de notre territoire pour nos agriculteurs de, enfin tous ceux qui ne comprendraient pas que les surfaces artificialisées ne soit pas pleinement mobilisés avant de les consommer du foncier disponible par ailleurs quant aux amendements pour le onze, l'article adopté en commission prévoit déjà la possibilité de recourir à une alternative au dispositif des ombrière cet amendement est donc satisfait une demande de retrait sinon défavorable le 180 contrairement à ce qu'affirment ces amendements, la notion de parcs de stationnement extérieur ne pose pas de difficultés d'interprétation, c'est donc un avis défavorable sur les 82 100 622 182 et 465 je partage l'intention de ces amendements, qui vise à exclure les parkings de poids-lourds de l'application de l'article onze nous avons en effet entendu dans le cadre des auditions que ces parkings pouvait connaître des contraintes techniques qu'on imagine bien, empêchant l'installation d'Brière je suis donc favorable aux amendements 182 et 465 qui exclut spécifiquement de l'application de l'article onze les parkings accueillant majoritairement des véhicules de plus de 7 tonnes et demie, je serai en revanche défavorable aux amendements 82 106 et 122 qui ne sont pas compatibles pour les 94 et 120 le fait de préciser que les parcs assujetties aux obligations de l'article onze doit être d'un seul tenant, ne me semble pas être une précision nécessaire je demande cependant sur ce point, l'avis du gouvernement sur le 435 ce sera un avis défavorable, c'est un moment qui visent à à revenir sur la porte de commission qui est proposé que la superficie soit, calcule en emplacement plutôt qu'en mètres carré pour faciliter l'application du dispositif pour le 298 ce sera un avis défavorable à cet amendement qui vise à abaisser le seuil d'obligation de 80 50 emplacements avec 80, nous avons souhaité rester au niveau d'ambition du texte initial car ce nombre d'emplacements correspond à environ carrés, même si il était évoqué son emplacement sur cette même surface donc un avis défavorable sur les 93 119 et 181 ce sera un avis défavorable, les airs parce que satisfait désert où s'effectuent les opérations de chargement et de déchargement ne sont par définition pas des emplacements au sens de l'article onze puisque ils ont une autre vocation Césaire seront donc décomptées dans la surface devant être couvertes par des ouvrières sur les 95 et 121 l'article adopté en commission prévoit la possibilité de recourir à une alternative au dispositif des hier pour autant que ces dispositifs alternatifs soit installé sur les mêmes entités foncière je savais même parc de stationnement changer cette formulation pour permettre la citation de dispositif alternatif sur l'unité foncière ne pourrait-il pas être une manière pour les personnes assujetties à l'article 11 échapper à leur obligation se prévalant, par exemple, des installations photovoltaïques qu'elles devront bientôt installé sur le bâtiment non résidentiel, je sollicite sur ce point, l'avis du gouvernement sur les 619 et 297 un avis défavorable à ces amendements qui retirent le pouvoir donner aux élus locaux dans l'application des dérogations à l'article 11 pour les 400 246 477 c'est un avis défavorable à ces amendements qui visent à prendre en compte les contraintes d'exploitation qu'elles peuvent être soumises les parkings notamment sur lorsque ceux-ci Servent accueillir des festivals, des circuits des fêtes foraines, je rappelle que l'obligation de couverture ne portera que sur la moitié de la surface des parkings qui met également que la mise en place dans prière n'empêche pas nécessairement la tenue de ces événements, même si ça peut compliquer dans certains cas, il faut le reconnaître, sur les 41 et 360 c'est un avis défavorable, changement d'affectation d'adaptation du service public me semble déjà couverts par la liste des critères permettant de déroger à l'obligation prévue par l'article onze notamment le critère permettant de déroger à l'obligation si les installations ne peuvent se faire dans des conditions économiquement acceptables, n'en rajoutons pas trop, car l'article onze serait illisible et inapplicable sur le 117 c'est un avis défavorable parce que satisfait en réalité parce que nous avons défini et je viens de l'évoquer à l'article 11 ce sont les élus locaux dans le cadre existant qui fixeront les dérogations donc il leur appartiendra d'exclure éventuellement les les sites que que vous évoquiez sur le 333 et 118 avis défavorable, la mise en place de dispositifs de perméabilité des sols n'empêche pas l'installation en mourir sur les parkings, ils ne font pas en faire un critère supplémentaire dans la liste de dérogations sur le 55 c'est un avis défavorable, il paraît difficile d'exclure à priori les parcs de stationnement qui n'ont pas vocation à être pérennisés, car il serait désartificialiser pour atteindre l'objectif de 0 artificialisation nette comment connaître 10 ou 20 ans à l'avance la liste des parcs qui devront être dans cette situation, je pense, en tout état de cause, qu'un parc qui a fait l'objet d'une d'un projet des artificialisation pourraient être couvert par la des dérogations dérogations prévues en cas de contraintes techniques sur le 255 c'est un avis défavorable, plutôt que supprimer le 8ème alinéa je propose un amendement 670 ce que j'ai développé de clarification de cet alinéa cet amendement précise que la possibilité, mais je l'ai, je l'ai expliqué tout à l'heure cinq cent sept 23 56 247 et 475 c'est un avis défavorable ne pense ne m'ont pas souhaité repousser les délais prévus par le projet de loi, ces délais sont réalistes, les repousser, c'est retarder d'autant plus le développement on fait confiance, bien sûr, à l'ensemble des accords pour être au rendez-vous de ses objectifs.

de couvrir les les parcs de stationnement extérieur mais qu'il y a des dérogations ces dérogations, elle s'applique aux parcs de stationnement extérieur lorsque des contraintes techniques de sécurité architectural ou patrimonial ne permettent pas d'installation des dispositifs. C'est le premier items, donc tout ce qui est poids-lourds et cetera et traités par ça, soit c'est un problème et on le fait pas, soit c'est pas un problème. Et on peut le faire, guillemets pour déroger, c'est lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiques. Acceptable, je le j'insiste sur ce point là, on ne peut pas opposer que ça serait très coûteux et que on fait peser une charge sur ce qui qui seraient amenés à respecter ses obligations puisqu'on on on suppose que l'on fait des opérations économiquement équilibré équilibré et, de fait, aujourd'hui, faire des panneaux photovoltaïques, c'est des opérations économiquement équilibrée, on peut imaginer à certains égards, qu'il y a des exceptions, et dans ce cas-là, il y a une dérogation. Et le 3ème élément, c'est un peu plus spécifiques lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie donc par rapport à ça c'est expliquera l'orientation de mes réponses

hop amendement pardon 82 c'est un avis défavorable 94 et 120 c'est donc avis du Gouvernement demandée par le le rapporteur, c'est effectivement un avis défavorable, il nous semble que la rédaction actuelle de l'article 11 qui vise les emplacements de parcs de stationnement pour l'application de l'obligation est suffisamment clair cette rédaction de porte pas à confusion quant au Champ d'application de l'actif amendement 435 je suis favorable, parce qu'il est clair que c'est plus facile de compter des mètres carrés que de compter des places, nous, on a compté des camions d'un compté plein de choses ces derniers temps, sincèrement content des mètres carrés, je pense que la sophistication de la rédaction, qui est sorti de la commission va rendre beaucoup moins facile, enfin

avis défavorable, hein c'est traité par le qu'il avait hâte sur la technique pour difficultés techniques, amendement 95 et 121 avis du Gouvernement demandées par la commission c'est un avis défavorable, le dispositif porté par l'article 11 vise à développer l'installation de procédures de procédés de production d'énergie renouvelable, sur des parcs de stationnement, parce qu'il s'agit de surfaces déjà artificiel artificialiser quand cela nous limitons la consommation nécessaire d'espaces naturels et l'artificialisation des sols votre amendement conduirait à reporter l'obligation d'équipements sur d'autres unités foncières pouvant naître pas artificialiser ou présentant des intérêts à préserver ce qui n'est ni dans l'esprit de la mesure, ni dans celle de la lutte contre l'artificialisation des sols 106 et 122 défavorable. le, qu'il avait hâte qui est prévu la dérogation prévue à l'article 11 permet de de couvrir ces situations et, au fond, tels que ces rédigé, c'est une façon de limiter la zone d'application, le périmètre d'application de la Loire, nous devons développer les énergies renouvelables on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible sur des parkings qui a accueil des camions, d'ailleurs c'est même dans certains cas. Plutôt venu nous disent les professionnels, amendement 182 et 465 défavorable, amendement 297 défavorable, amendement 619 favorable parce qu'il nous semble que la rédaction qui était initial était plus précise et de nature à préserver les contentieux des contentieux, les décisions qui seraient prises en vertu de cet article, amendement 400 défavorable, amendement 246 et 477 défavorable puisque les cas d'exemption comprend également les contraintes techniques d'exploitation oui c'est déjà couvert satisfait amendement 41 et 367 défavorables, amendement 117 favorable, il nous semble que la rédaction permet de clarifier et de protéger juridiquement l'application de ce texte, de limiter les contentieux, amendement 333 défavorable, amendement 55 défavorable, défavorable, amendement 118 défavorable là je rejoins, je pense, pour l'essentiel les réponses du rapporteur, amendement 255 favorable, favorable, pourquoi l'amendement vise à supprimer la disposition tendant à une répartition par les communes des ombres hier sur l'ensemble des parcs de stationnement en tête, en effet, telle que rédigée cette disposition qui qui a été introduite par la commission est inapplicable, il est impossible de mutualiser les obligations d'installation de bruyère entre des propriétaires ou gestionnaires de parkings extérieurs différents qui peuvent par ailleurs être des personnes privées ou publiques différentes amendement 670 défavorable pour les mêmes raisons, amendement 605 défavorable et là je vais reconverti G avec les avis du rapporteur, donc 107 défavorable et de 123 et 56 247 et 475 défavorable, ce sont tous les amendements de report de l'application de l'article. Bien, merci, donc nous avons l'ensemble des avis je les redonnerai au fur et à mesure de des des votes, monsieur le rapporteur. monsieur le président je souhaiterais simplement préciser parce avant le le le vote que je je suivrai l'avis du gouvernement, assure à chaque fois que je l'ai demandé sur certains amendements et puis compte tenu de la position du gouvernement sur l'amendement 117 de notre collègue Cédric je prends sur moi, parce qu'on évidemment je vais revenir sur une décision de la commission mais je proposerai de changer mon avis le transforme en avis favorable. Oui pour dire que je retire les amendements 93 et 94 ont effectivement, j'ai compris qu'ils étaient satisfait enfin en tout cas les propos de la miss viendront levé tous les doutes qui pouvaient subsister juste sur l'amendement 95, j'ai l'impression qu'il y a une erreur d'interprétation et je voudrais pas qu'on croit, ici, que l'ensemble des cosignataires de ces amendements veulent artificialiser des zones qui ne le sont pas, en transposant l'installation des panneaux photovoltaïques qui étaient prévus sur les aires de stationnement sur d'autres endroits, c'est absolument pas ce que dit cet amendement et je pense que l'exposé des motifs, est très clair, il dit juste qu'il cherche à faire des installations de production d'énergie renouvelable au mur hier, coût pour la collectivité, en permettant que l'obligation de production qui est liée à la surface de stationnement puisse être réalisée sur un autre bâtiment doté propriétaire le même gestionnaire qui est situé sur la même unité foncière, il dit uniquement ça et l'autorise à faire en sorte que cette production elle puisse au lieu que ce soit des panneaux solaires, on peut très bien imaginer des ballons d'eau chaude, si dans le cycle industriel qui a lieu sur cette unité foncière, on a un enfin voilà, c'était juste pour corriger les propos de la Ministre parce que j'ai eu l'impression qu'on nous on va, on nous indiquait qu'on était prêt à recouvrir des champs pour ne permettent de panneaux solaires sur un Parking, ce qui était absolument pas ce qui a été visé par cet amendement et donc je vais le maintenir. Merci monsieur Corbizet. par rapport à l'avis favorable du gouvernement parce que donc notre excellent rapporteur reviendra sur l'amendement 255 puisqu'au départ il avait mis un avis défavorable et que le con, le gouvernement a émis un avis favorable compte tenu de la précision juridique a porté l'amendement de mon collègue Cabanel. remercie Monsieur Pointereau. l'amendement numéro 11 rectifié bis de Madame May puisque apparemment il est satisfait, moi je me réjouis de de voir qu'on va pouvoir mettre du photovoltaïque sur toutes ces ces parkings de grandes surfaces, notamment, qui qui vont permettre de faire de l'énergie renouvelable, mais moi je me pose une question, et je la pose à Madame la Ministre, qui a été ministre de l'Industrie, quelle est la part et je rejoins les propos de mon collègue Cédric Vial, quelle est la part de ce qui peut être produit en France, en terme de panneaux photovoltaïques, parce que j'ai l'impression quand même que toute l'Asie, et particulièrement la Chine doit se réjouir ce matin de de voir qu'on va mettre des peut-être des, des milliers d'hectares de de photovoltaïque qui vont être produits en Chine, en Malaisie, aux Philippines et je crois que notre balance du commerce extérieur va en prendre encore un sacré coup.

ce projet de loi a des intentions qui sont tout à fait intéressante mais mais considérer que c'est l'urbanisme ou l'autorisation qui fait le qui fait le projet, c'est, c'est une erreur, il y a évidemment la filière, il y a évidemment d'autres enjeux qui aurait dû me semble-t-il, a traité, traité en en parallèle mais on y reviendra peut-être, j'ai j'ai une question à vous poser à tous les deux monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, parce que je j'ai encore un doute, même si j'ai entendu un certain nombre d'éclaircissements et je vous remercie par contre aussi sur le la l'amendement 117 j'ai un doute pour savoir à quoi s'appliquent cet article de loi et quand le législateur n'est pas clair, c'est le juge qui décide et je préférerais qu'on soit clair ici dans cet hémicycle, sur la définition d'un Parking extérieur puisque vous me dites, il y a pas de problème de définition non aujourd'hui le code de la voirie routière alors je l'ai pas sous la main mais le code de la voirie routière donne une définition qui n'est pas celle dont on parle donc, soit on est sûr de nous, et à ce moment-là, effectivement, c'est le juge qui décidera si une haute définition ou celle qu'on a en tête aujourd'hui quand on vote et la bonne, ou alors c'est lui qui sera peut être que pour l'esprit de la loi et pour dans le dans le cadre des jurisprudences ultérieures, il serait utile prenne 2 minutes que vous preniez 2000 pour pour clarifier ce qu'est un parking extérieur par rapport à une aire de stationnement extérieur je vous dis aujourd'hui le le le code de la voirie ne dit pas exactement ce ce ce dont on a discuté dans cet hémicycle, donc je pense que ça vaudrait le coup quand même qu'on dit est-ce qu'un Parking de supermarché, un Parking gratuit extérieur

Merci Monsieur Dantec. d'un quand même un peu. Quand même un peu mais mais je présume que c'est juste une interrogation c'est : c'est pour ma culture personnelle, on est bien d'accord que personne ici au moment de Noël ne met au pied du sapin hein jouets fabriqués en Chine, parce que pour les jouer, c'est 57 pour 100 les jouets achetés en France qui sont fabriqués en Chine, c'est plusieurs milliards sur la feuille sur la filière photovoltaïque, la part de valeurs liées à la Chine est relativement enfin parce que il y a l'installation il y a même, je vous le rappelle, des filières en France le président Gontard, il est particulièrement attentif, il y a même une entreprise en Loire-Atlantique, qui fabrique des panneaux photovoltaïques, alors même si je suis d'accord pour dire qu'il faut structurer la filière, il n'y a que sur le photovoltaïque, qu'on a un tel débat alors que sur des dépenses autre on n'a absolument pas la même monté au créneau, donc moi je m'interroge : pourquoi toujours ce 2 poids, 2 mesures, même si on est tous d'accord pour dire qu'il faut une filière en France mais j'espère que personne à Noël achètera des jouets fabriqués en Chine.

Merci monsieur le président, pour ceux qui chercheraient des idées de cadeaux à Noël, au-delà de l'achat d'un panneau photovoltaïque je vous incite à acheter du Charolais de la viande charolaise ou du vin de Bourgogne qui sont produits en France, monsieur le président je vais annoncer le le retrait. Je vais annoncer le retrait de l'amendement 400 puisque j'ai entendu dans la bouche de la ministre que les contraintes techniques qui pouvait être retenue comme dérogation pouvait être, d'après ce que j'ai compris, donc, des contraintes techniques de structures mais également des contraintes techniques d'exploitation et à partir du moment où il sera gravé dans le débat parlementaire que par contrainte technique, il faut aussi entendre contraintes techniques d'exploitation naturellement l'amendement perd de son intérêt, j'en profiterai tout de même pour interroger la la ministre sur le une interrogation qui est la mienne, on commence à à voir apparaître un certain nombre de prototypes de véhicules électriques qui sont capables de recharger leurs batteries grâce à l'énergie solaire directement et donc je suis saisi à cet instant d'une interrogation : si vous mettez des ombres hier sur tous les parkings, comment pourrons-nous assurer la recharge de ces véhicules en stationnement, si vous voulez, privé de soleil. Madame Nandor. Merci monsieur le président, je voulais juste dire que la France a du savoir-faire pour la production de de panneaux photovoltaïques, il y a une reprise réunionnaise qui produit depuis de nombreuses années des panneaux photovoltaïques, et qui est aussi installé aux États-Unis, il me semble que mon collègue à visiter cette entreprise il y a du savoir- faire français dans le domaine des énergies renouvelables et de la construction des panneaux photovoltaïques et j'y crois.

de la possibilité d'accorder des délais supplémentaires en cas de difficultés d'approvisionnement, donc je ne sais pas si c'est le moment de faire le débat tout de suite sur la nécessité de de se doter et d'encourager et de stimuler la filière française mais j'espère que Madame la ministre, nous donnera des des réponses tout à l'heure. Bien, merci, donc encore une prise de parole Monsieur Salmon. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, je reviens en 2 mots sur la filière effectivement c'est regrettable que nous n'ayons pas une filière française, on a même pas vraiment une filière européenne j'ai entendu Madame la Ministre, la première ministre, l'autre jour, lors du débat sur la politique énergétique de la France s'engager sur sa volonté de mettre en place une filière française, donc je sais pas si vous avez Madame les ministres des des éléments sur ce sujet, ce que l'on sait, c'est que dans les 20 années à venir, on va devoir installer à peu près 3 à 5 gigawatts par an donc c'est dans les 20 années si il y a une vraie volonté de mettre en place une filière, il n'est jamais trop tard, on peut y aller et je pense qu'il faut être très volontariste dans ce sujet. Oui, merci Monsieur le Président, je souhaite intervenir sur ce point, mais un peu plus tard, mais compte tenu que le débat est lancé, je, je vais le faire à cet instant. Nous devrons être très attentif. à l'appel d'air que nous allons. Ouvrir. Avec les décisions que nous sommes en train de prendre. Je vais vous parler d'un peu d'expérience. Et vous pourrez contrôler mon propos. Le début du photovoltaïque, mais c'est le début de toute opération 5, pareil pour l'éolien dès lors que vous lancez et que vous garantissez un certain niveau de. Vous Vous avez un appel d'air sur le marché qui fait que le prix de vente du produit. N'est pas dans le Champ concurrentiel. Et si je reprends l'exemple du photo-voltaïque pour l'avoir vécu, ceux qui ont investi à 14 ans. Regardez le prix qu'ils ont payé au mètre carré. Et dès lors que le prix d'achat a baissé soudainement.

entre le moment où le prix d'achat été modifié, il a été divisé par 2, aujourd'hui, est divisé par 3, là il y a eu des améliorations techniques, mais en l'espace d'un an, la division par 2, économiquement, il ne faut pas nous l'affaire. je, j'évoque ce point là parce qu'il ne s'agirait pas. Et, et c'est pas un propos de, de remise en cause, hein, je ne peux pas le prendre dans cet angle-là, mais je j'alerte à cet instant là et il faudra qu'au niveau de la concurrence soit assez actif parce que sincèrement, on donne des raisons vraiment d'espérance et de marché offert hélas à beaucoup de pays en dehors de notre territoire national ou voire européens et, effectivement, lorsque certains parlaient de bilan carbone et c'est le Sénat qui l'a introduit dans un dernier texte il y a le prix mais il y a aussi le bilan carbone noir, soyons attentifs. Merci, cher collègue, monsieur le président Gontard. Merci monsieur le président, je ne pensais pas non plus intervenir sur la question de la filière, mais puisque du coup, il y a le le débat et puis on pourrait revenir tout tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même central est important et c'est vrai que pour le coup, on a peu d'indications et peu d'éléments sur ce texte sur cette question de la sur c'est sûr que les projections sur les 20 ans en termes d'installation de panneaux photovoltaïques ont enfin je pense qu'on a aucun secteur où on a un avenir, comme ça il y a la question effectivement concurrentiel mais à la question : carbone, on aura des amendements d'ailleurs sur comment, justement dans la commande publique on intègre réellement cette question là, il y a une question européenne c'est, c'est évident, mais actuellement je pense qu'il faut quand même qu'on sache que, en France, non seulement on a du silicium et on sait le fabriquer, on sait le faire, la situation actuelle, c'est que on a fermé une unité en Savoie notamment qui fabriquait du Silicium hein, le groupe Ferro globe et l'entreprise fait Open, donc on est quand même dans cette situation là, on a encore une entreprise en Isère, qui fabrique du fait et qui fabrique du du silicium et qui est capable justement de fournir pour les panneaux photovoltaïques qui est en grande difficulté, je sais que Madame le Ministre, connaît très bien le le sujet, j'étais la semaine dernière à Photowatt, la seule entreprise française qui fabriqué

on a pris des photos, on a pu la visiter fonctionnent plus et ce qui nous disait c'est qu'il y a une vraie question sur à la fois le savoir-faire sur les compétences qu'on a des machines maintenant qu'on a achetée en Allemagne pour ses fabrications là maintenant qu'on ne trouve plus qu'en Chine, puisque tout le savoir-faire est parti en Chine et qu'on devient complètement dépendants de la Chine, même sur la fabrication de ces machines, donc il y a une vraie question à se poser, et là je pense que la volonté politique à une véritable importance. Merci beaucoup, alors je veux juste d'abord faire une précision sur l'amendement 11. Parce que je ne pense pas que le texte actuel le satisfait Honnêteté intellectuelle sur les autres oui sur l'amendement 11 spécifiquement, il me semble que non sur je vous donne mon point de vue du gouvernement, c'est pour être carré sur la question des des filières industrielles, je pense que c'est un très bon débat, c'est un très bon débat puisque, effectivement, se pose la question de quelle visibilité on donne au marché quelle stabilité on donne au marché qu'elle compétitivité ou les fabrications françaises et européennes, s'agissant des panneaux photovoltaïques, alors déjà en moyenne je vais reprendre le propos de monsieur le sénateur Dantec, vous savez qu'en France, pour un Euro, ou pour 100 euros dépensés 36 heures Euro le sont par de la fabrication française 64 euros par la fabrication étrangère donc ce n'est pas un sujet qui est propre à la fabrication des des énergies renouvelables, c'est un sujet plus structurant de réindustrialisation sur lequel le gouvernement est engagé depuis plusieurs années et dont le point je dirais central et la question de la compétitivité relative de la France par rapport à d'autres pays et qui a amené à proposer un certain nombre de mesures pour augmenter l'attractivité du site France par rapport à à ses concurrents européens et à ses concurrents extra-européens où ça, c'est une discussion qui nous emmènerait très loin si maintenant je reviens au sujet des des filières énergies renouvelables, vous le savez, ce sont des filières qui sont aujourd'hui accompagnés dans France 2030 au-delà de ce que nous avons pu porter avec Bruno Lemaire, notamment sur la filière hydrogène sur la bas carbone sur la filière batterie électrique avec 3 sites de production dans le nord et dans le le qui allait et toute une vallée européenne de la batterie qui est en train de s'installer là-bas sur l'investissement que nous avons lancé dans France 2030 avec plusieurs appels à projets qui couvre les différentes filières que que vous mentionnez mais vous avez raison de souligner qu'en terme d'équipements, je parle pas effectivement de tout ce qui entoure l'installation de génie civil, l'ingénierie, les bureaux d'étude parce que effectivement ça c'est c'est du service autour des énergies renouvelables et ça crée de la valeur en France, en terme d'équipements, force est de constater que sur. Les panneaux photovoltaïques, c'est pas un grand succès, on a pu constater quand. 3 ans, marché chinois à inonder l'Europe ben qui a particulier à la France à inonder l'Europe et qu'on doit avoir à peu près plus de 80 % si ce n'est 90 % de panneaux photovoltaïques d'origine asiatique, par rapport à ça. Il y a 2 actions il y a une première action qui consiste à avoir des panneaux photovoltaïques voltaïque qui soit. Compétitifs et produit de manière industrielle, parce qu'il est une question de quelle quantité et il y a une 2ème, action qui consiste également à voir dans les cahiers, les appels d'offres des définitions environnementales environnementales qui englobe donc la question de la logistique des critères environnementaux, voire des critères de fabriquer en Europe qui soit plus sérieux ou plus, on va dire, exigeant, vous savez que, à mon initiative, les codes, les cahiers des charges administratives générales prévoit qu'il y a automatiquement automatiquement une clause environnementale dans les marchés publics, automatiquement, après, on peut s'en écarter, c'est le choix de l'acheteur public mais je pense que pour les communes pour les acheteurs publics cette clause est vraiment intéressante effectivement pour accorder à la fois vision industrielle et visions environnementales et éviter d'importer des émissions carbone, de l'autre bout du monde, ça c'est, c'est c'est un point important, au-delà il faut renforcer la filière renforcer la filière c'est ce que nous faisons avec France 2030 et il faut au niveau européen à avoir des actions communes, et vous savez que à Thierry Breton vient d'annoncer une alliance européenne du solaire, avec des investissements pour justement rebâtir cette filière, on part de loin, je ne vais pas mentir devant la représentation nationale, mais je trouve que cette discussion est très intéressante parce qu'on va l'avoir bientôt sur les éoliennes marines.

cette motivation à donner de la visibilité à une filière industrielle à porter des sites industriels, sur le territoire et à permettre à ces sites de s'est développé avec des marchés français soient pris en compte et qu'on est bien en tête les 6500 emplois Directs et je ne parle pas des indirect, mais vous savez que c'est fois 3 fois, 4 dans le monde industriel de cette filière éolienne marine je vous remercie.

je vais le conserver, parce que je pense qu'il est important puisqu'on propose de faire au moins la moitié en en panneaux photovoltaïques sur les parkings, mais l'autre moitié de faire en sorte que le terrain ne soit pas imperméable et qu'on qu'on végétalisées, donc ça va dans le sens aussi de de l'environnement et de des de la non-artificialisation des des sols donc je je conserve. Bien, merci, cher collègue, donc nous allons procéder au vote ah avant chaque article je vais rappeler les avis qui ont été données. Et si quelqu'un souhaite retirer l'amendement à l'instant où j'ai non serait son numéro. Qu'ils se manifestent aussitôt ce qui nous évitera de multiplier des votes inutile donc. L'amendement numéro 11 donc est maintenu avec un double avis défavorable qui est pour. je viens de dire que l'amendement était maintenu avec un double avis défavorable. Donc, l'amendement est maintenu avec un double avis défavorable et donc je le soumet au vote qui est pour. C'est.

je le retire, président le 82 rectifié double avis défavorable. Il est maintenu,

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 298 avec un double avis défavorable qui est pour.

Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Le son 21 même vote le 106 rectifié

même vote le 182 rectifié : avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, le 465 rectifié même vote. Le 297 amendement de Monsieur dont avec double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 619 rectifié : avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 400 rectifier retirer le 246 et qu'un double avis défavorable. Retirer le 200 le 477 pardon avec un double avis défavorable, il est maintenu, retirer le 41 rectifié avec un double avis défavorable maintenue oui maintenu, donc il est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 367 rectifié qu'un double même vote le 117 rectifié avec un double avis favorable.

Retirer le 255 avec un avis défavorable de la commission. Favorable du gouvernement Monsieur Corbizet. Dans incapacité le revirement de mon rapporteur merci. Donc je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Je pense qu'il est adopté. Six cent 70. Tombe. L'amendement 605 rectifier avec un double avis défavorable,

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 400 rectifier il est identique, donc même votre vote le 56 rectifié Monsieur Vial vous le maintenez double avis défavorable. Oui, maintenu donc qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 247 même vote et le 475. Identique. Bien, nous avons donc terminé avec ses trente-six amendements en discussion commune nous poursuivons avec l'amendement 609 rectifié madame avait. Cet amendement propose, sur la base des modifications opérées par la commission de prendre en compte la notion d'emplacement et de l'adapter aux zones non internautes connectés en portant l'obligation d'équipement des parcs de stationnement extérieur existants en nombre hier photovoltaïque à 40 emplacements. Il la commission. Je demande l'avis du gouvernement, j'entends bien les préoccupations et je souhaite avoir travaillé, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Alors ce sera une demande de retrait votre amendement vise à. Prévoir un seuil d'âge assujettissement à l'obligation de réaliser des hier des 40 emplacements pour les parcs situés dans des zones qui ne sont pas interconnectés le dispositif porté par l'article 11 traduit un équilibre entre ambitions énergétiques, environnementales et contrainte pour les assujettis les seuils doivent être fixés dans une perspective de faisabilité technique et de rentabilité économique, c'est tout le la logique votre amendement s'il était adopté, serait de nature à compromettre cet équilibre, et donc l'efficience du dispositif retrait ou avis défavorable.

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues se prêt cet amendement vise à calculer le taux de couverture d'dont Brière photovoltaïque en tenant compte de la surface totale des parcs de stationnement extérieur géré par une un exploitant aéroportuaire, et non de la surface parc par Park, en tout état de cause au moins la moitié de la superficie globale des parkings extérieurs des aéroports devraient être équipés d'ombrière photovoltaïque, ainsi que le dispositif favorisant la perméabilité l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur le plan financier, les coûts de raccordement au réseau, qui représentent entre 5 et 15 % de l'investissement total serait pénalisant en cas de multiplication de parking extérieur et qui perdent en Brière, un autre les parcs de stationnement de grandes superficies permettent des économies d'échelle et une rentabilité plus élevée de l'investissement, c'est pourquoi le cas spécifique des aéroports dans le cas spécifique de l'aéroport, il est proposé de couvrir Brière en grande partie voir en totalité la superficie de certains parkings extérieurs, tandis que le taux de couverture d'autres parkings extérieurs dans l'emprise de l'aéroport sera inférieur à 50 % même si leur superficie dépasse les 2500 mètres carrés, je vous remercie. Merci l'amendement 467 monsieur Moga. Merci monsieur le président, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, mon amendement comme celui que viennent de présenter notre collègue Stéphane Sautarel étonnamment demande de bon sens, il consiste à apprécier le pourcentage de couverture sur la le sable des parkings de l'aéroport et non de Parking par Parking. Merci l'amendement suivant le 366 Madame Dindar. Oui, monsieur le président merci, il me semble que cet amendement est défendu déjà par ceux présentés par mes deux collègues. 368 c'est vous aussi Madame Dindar celui qui suit. Bien, merci, ensuite, 2 amendements identiques monsieur Cabanel 248. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement a pour objectif d'adapter les obligations aussitôt qui dispose de plusieurs parcs de stationnement extérieur ce cas particulier peut notamment concerner les sites événementiels d'expositions ou de congrès dans ce cadre, il semble plus pertinent de prendre en compte l'ensemble de la surface des parcs de stationnement, plutôt que de considérer chaque part de stationnement séparément le présent amendement propose donc d'accorder plus de souplesse, le gestionnaire des parcs de stationnement, hein, permettant d'apprécier l'obligation d'équipements photovoltaïque à l'échelle du site. Mathieu Genêt pour un amendement identique. Oui, Monsieur le Président, encouragée par le président Karoutchi je souhaite prendre la parole pour appuyer la défense qui vient d'être faite de cet excellent amendement déposé par notre collègue Boccuillaut Fontimp j'en profiterai également pour appeler à nouveau l'attention de la Ministre sur la question que j'ai posée tout à l'heure sur les véhicules qui pourrait éventuellement se recharger seul et au-delà de c'était pas un trait d'humour, c'est une vraie interrogation pour comprendre comment vous pilotez la transition énergétique au niveau du ministère est-ce que vous intégrez ce type d'évolution technique pour ne pas être en retard d'une d'une évolution technologique, merci de votre réponse. Merci, monsieur le rapporteur, avis sur ces six amendements en discussion. Je vais donner un avis Farab l'sur 2 de ces amendements, et en particulier donc précisément 248 et le 476 ils permettent de mesurer le respect de l'obligation à à l'échelle d'un site regroupant plusieurs parcs de ça sûrement extérieur, c'est du bon sens, ce sera donc un avis favorable pour ces 2 un un avis défavorable, par conséquent, au 44 167 et 368 qui sont, de fait, satisfait, puisqu'il prévoit un dispositif analogue de répartition pour les plateformes aéroportuaires et puis enfin un avis défavorable sur 366 aucune raison que l'obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement des aéroports, si d'autres surfaces sont disponible pour installer des procédés de production d'énergie renouvelable, donc l'obligation soit senti satisfaite. je vais donner un avis défavorable à l'ensemble des amendements mais j'ai déjà expliqué les motifs et donc ça me laisse 30 secondes pour répondre à la question sur les véhicules, les véhicules qui peuvent se recharger seul s'agissant de de ces véhicules tels qu'est construit, aujourd'hui l'obligation de couvrir les parkings, je rappelle que c'est une. Obligation pour la moitié de des parkings, ce qui laisse l'opportunité pour l'autre moitié d'accueillir des véhicules électriques et compte tenu de l'équipement que nous lançons aujourd'hui en véhicules électriques et il semblerait que ce soit tout à fait équilibré à horizon 2035 voilà et s'agissant de de quelle manière on intègre ces technologies dans les stratégies de de décarbonation

un peu frustre, hein, compte tenu de tout ce qu'on doit faire tourner sur la stratégie nationale bas-carbone mais qui nous permettre d'avoir des des idées des des grandeurs et de vérifier que l'ensemble de nos, de nos trajectoires boucle ou ne boucle pas et où sont les les impasses, c'est comme ça que nous procédons donc on sait qu'il y a un certain nombre de technologies qui vont avoir leur usage propre, on n'a pas aujourd'hui une notion de quelle sera la technologie qui, entre guillemets, gagnera je j'ai dans un autre contexte par, par exemple, parler du véhicule tout, qui est également dans la le travail que nous faisons sur la décarbonation, un point intéressant c'est évidemment pas des sujets qui impacteront avant 2030, hein, faire des trajectoires raisonnablement robuste jusqu'à grosso modo 2030 et 2, essayer de faire preuve d'autant que possible de neutralité technologique, c'est pas toujours évident pour éviter d'injurier l'avenir est passé à côté d'une technologie qui va s'accélérer, qui sera la technologie gagnante et nous avons une révision tous les 5 ans de nos trajectoires.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 467 rectifié présenté par Monsieur Moga double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 366 rectifié présenté par Madame Dindar double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 368 Madame Dindar même vote n'est pas adopté et le 248 rectifié et le 476 qui sont identiques, avec un avis défavorable du gouvernement est favorable de la commission, donc il est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés ensuite le 83 rectifié monsieur

Fillon le présent article crée des nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieur qui devront être équipés d'Ombrie à photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface des emplacements de stationnement donc le présent amendement propose de désigner le propriétaire du parc de stationnement en tant que débiteur de ses obligations la responsabilité lui incombant : de fait, même si, dans ces différents cas de figure, c'est une fini le propriétaire qui est compétent, responsable il semble utile de clarifier cela dans la nouvelle rédaction. Monsieur le président, je comprends bien l'intention de cet amendement qui vise à faire porter la responsabilité de l'application de cet article onze sur le propriétaire d'un parc de stationnement, plutôt que sur son gestionnaire, toutefois je ne mesure pas totalement les implications que cela pourrait avoir, notamment pour les collectivités territoriales dans le cadre de DSP de leur parc de stationnement, gérée par des tiers, donc je demande l'avis du gouvernement. Alors, peut être une précision pour pourquoi avoir utilisé ce terme de gestionnaire, parce qu'il permet de faire supporter le coût de la mise en conformité avec les obligations par la personne tirant directement un bénéfice de l'exploitation du parc de stationnement si le parc est géré par un tiers, c'est donc lui qui doit supporter l'obligation prévue qui sera compensé par les revenus de l'installation, si le parc n'est pas géré par un tiers mais directement par son propriétaire, c'est bien ce dernier qui assumera l'obligation fixée par cet article. Du coup, je pense que le terme utilisé dans l'article, plus précis, puisqu'il est moins réducteur que celui de propriétaire. Bien donc une demande de retrait il est retiré.

donc c'est déjà, je dirais, hein, un amendement un petit peu défaitiste c'est un amendement d'appel dans le sens où on aimerait, Madame la Ministre, vous avez répondu sur l'éolien Offshore et et on aura l'occasion d'en reparler sur l'article 12 et et je rejoins complètement votre argumentaire sur le fait qu'il existe dans ce domaine une une filière française qui est puissante qui s'est implantée avec l'appui des collectivités locales, malheureusement dans le domaine du photovoltaïque, on en est loin, quels sont les moyens véritablement dont la France se donne pour développer une filière française du photovoltaïque, c'est l'objet de cet amendement d'appel plutôt que de battre en retraite et en disant, ben oui, on admet des rollers, des des retards parce que parce qu'on ne saura pas fournir. la vie. Défavorable de la commission cet amendement qui supprimerait un apport de bon sens, adoptée par notre commission et celle des affaires économiques, d'ailleurs, donc c'est un avis défavorable. Ah, de Madame la Ministre. d'un certain nombre de composants d'équipements, on l'a vu sur la filière automobile récemment avec l'école, les semi-conducteurs, donc oui, il faut développer une filière de photovoltaïque, il faut qu'elle soit compétitive, il faut a minima, qu'elles soient européenne, si ce n'est française et c'est tout l'enjeu de l'Alliance européenne solaire qui a lancé le commissaire breton, mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain, néanmoins, dans l'attente, il ne faut pas retarder la mise en oeuvre de la décarbonation de notre économie et je veux redire ici que cette question de l'empreinte carbone, elle est transversale à tous les secteurs, elle est transversale à tous les secteurs, elle doit nous amener à avoir des décisions industrielles fortes, ce que nous essayons de faire depuis 6 ans, 5 ans maintenant, mais elle n'est pas propre au secteur des énergies renouvelables et donc il faut avoir la même vigilance et exigence dans tous les secteurs, y compris les jouets. c'est, c'est juste pour ajouter une Pierre au au débat qui vient, qui vient d'être lancée sur la filière photovoltaïque, je pense qu'on est tous conscient ici des enjeux de du développement de cette filière qu'on se donne, qu'on puisse se donner les moyens plutôt que des incantations pour pour y arriver, je viens d'un département, la Savoie où vous connaissez probablement Madame la ministre est implantée l'INS, l'Institut national de l'énergie solaire qui a été précurseur sur le sujet et à proximité Monsieur Gontard, l'a dit tout à l'heure, nous avions une entreprise Photowatt à Bourgoin-Jallieu qui qui produisait, qui est en difficulté depuis un certain nombre d'années et et et et pour les, pour lesquels on a besoin d'un appui et on a besoin d'un appui pour cette entreprise comme pour d'autres qui qui ne peuvent pas relever de la simple incantation la filière silicium, ça a été dit aussi tout à l'heure, on avait une entreprise là la seule productrice de de de silicium en France et en Europe, le gouvernement a été absent au moment de la fermeture de de ce site, absent, Madame la Ministre, aucune solution n'a été trouvée pour pour permettre au et le la reprise de ce site qui est toujours en friche,

en 3 ans ou en 5 ans, c'est pas le temps nécessaire pour créer une filière française, donc on sera forcément dépendant non pas 34 % ou à 60 % à 100 pour 100 de de d'approvisionnement étrangers et on a besoin de temps et on a besoin de lisibilité et quand tu l'obligation et sur une période aussi courte on ne n'offrent pas de, de, de visibilité à une industrie qu'on voudrait structurer et mettre en place et donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, autant l'incantation est importante, le le le le souhait que politique, on affirme tout c'est important, par contre, il y a un vrai enjeu politique pour développer ces filières, aussi bien sur la production que sur le retraitement de du photovoltaïque. Merci, cher collègue, donc nous allons passer au au, Madame la Ministre. Voudrait dire que les un milliard d'euros qui sont dans France 2030 et qui ont de l'EI lieu à trois appels à projets pour soutenir les différentes filières d'énergies renouvelables, c'est pas tout à fait de l'incantation, les 9 milliards d'euros qui sont investis sur l'hydrogène bas-carbone c'est pas tout à fait Limp quant à Sion ces 10 projets de futures usines qui sont d'ores et déjà financés et soutenus par le gouvernement français, donc je peux pas laisser dire ça et s'agissant de faire Open, je rappelle qu'il y avait 6 sites qui risquait de fermer six en France, qu'on en a sauvé 5 et qu'on a sauvé toutes les productions, c'est-à-dire il y a des reports de production de différentes qualités de silicium sur les 5 autres sites et un des leviers d'ailleurs, c'est toujours intéressant la politique énergétique un des leviers qui a permis de sauver faire Open, c'est la reine toujours intéressant à noter.

On parle de la construction, mais il faut aussi parler de la déconstruction. Les premiers panneaux photovoltaïques ont été installés sur notre territoire. à ce que je sache, on ne sait pas les déconstruire. alors, quand on imagine un investissement, il faut penser aussi à la fin de cet investissement. Et autant nous devons avoir le souci de produire sur notre territoire, autant nous devons avoir le souci en fin de vie, comment nous recyclons et ceux qui sont recyclables et dans quelles conditions nous allons le faire au niveau de cette énergie, je crois que c'est essentiel parce que personne ne l'aborde, or on sait, je répète : les premiers panneaux photovoltaïques, aujourd'hui on ne sait pas les déconstruire, on a tous en souvenir, hein, un sujet dont on reparlera tout à l'heure, c'est de l'amiante. Au début, on a tous et, aujourd'hui, qui se retrouvent dans la panade avec les plaques de fibro amiantés et cetera et donc c'est un sujet qu'il faut aborder dès sa construction. Président Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, je juste sur quand même le, le fait de pouvoir recycler les panneaux, on sait très bien le faire actuellement, et même sur les anciens, donc le Silicium on sait, on sait à peu près faire mais pour revenir sur ce qui a été dit sur la question de la la filière et sur la filière dans son ensemble effectivement était parler de faire Open avec avec le Silicium Madame la Ministre, moi j'entends à chaque fois vous nous dites, il y a plusieurs milliards qui sont faits pour de nouvelles

aussi conforter des sites de production qui, eux, sont très gourmands en carbone, notamment avec l'utilisation du du charbon, alors que, en France, on a l'utilisation de l'hydroélectricité et donc avec une solution, une solution décarbonnées donc je pense que ça c'est important de regarder ça et puis ensuite sur la volonté politique,

donc l'État a quand même des choses un petit peu à dire, on a un projet, un très gros projets photovoltaïques sur l'ancienne site nucléaire de Creys-Malville 26000 panneaux ont été installés, c'est juste à côté, quel choix a été fait par EDF, puisque c'est un projet EDF bah, c'est de ne pas utiliser les panneaux de sa filiale alors qu'il pouvait totalement le faire, notamment via les les marchés, les marchés publics, ils ont fait le choix de choisir des panneaux, des panneaux chinois, donc là oui, il y a une volonté politique et là oui, vous avez la main à travers EDF, surtout si en plus le capital passe à à 100 pour 100, donc je pense que là il y a vraiment matière à agir et agir rapidement et ne pas repousser sur de nouvelles installations en permanence. Merci Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président, en complément de ce qu'a dit Madame la mini-je crois que on est sur un débat important du con là maintenant et on aura moins tout à l'heure donc, c'était important de le tenir bon, moi je suis tout à fait d'accord avec Daniel Gremillet, il faut prévoir les filières de recyclage tout de suite, mais comme l'a dit le président Gontard, c'est le cas sur le photovoltaïque, parce que moi je l'expérience dans mon département natal du Finistère, on n'a pas fait de REP sur la filière graphite-gaz du nucléaire on est le bec dans l'eau, on sait pas la déconstruire, elle reste au milieu, 35 ans après on sait même pas percer le coeur du réacteur, donc oui il faut des filières de démantèlement des productions d'énergie électrique, on est bien d'accord, ensuite, il me semble que, on doit faire preuve effectivement de de prospective, il y a madame la ministre a parlé du film fortifie

ce qu'on ne dit pas, c'est que le film forcé qu'il faille européen, c'est ce qui va permettre à l'OMC, de mettre des taxes carbone aux frontières, si on n'a pas le fil forfait il faille on ne peut pas l'OMC maître de taxe carbone aux frontières et c'est cette taxe carbone aux frontières qui va permettre aussi de remettre dans le coût des importations, le coût carbone et notamment les panneaux chinois ont un coût carbone. Bien plus important que les panneaux qu'on fabrique chez nous, donc avec la taxe carbone aux frontières nos panneaux redevienne compétitif et ça je crois qu'il faut l'avoir en tête dans la mise en oeuvre dès maintenant de cette filière qui sera demain compétitive à partir de là, et ça je trouve que on ne fait pas le lien parce que j'entends, même des fois sur les bancs le fait dire : on fait un effort démesuré qui va nous affaiblir non cet effort de réduction des émissions, c'est ce qui va nous rendre plus compétitifs sur le marché français et européen de demain, donc ça me semblait important de le dire, et en trois secondes ne donnait pas de bouteille de Bourgogne, même si c'est très bon à vos enfants à Noël. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, bon ben c'est bien cet amendement du groupe socialiste permet qu'on parle d'une question de la filière industrielle. Puisque, depuis hier, on a un débat mais on on évite un certain nombre de sujets dont la filière industrielle. Non, mais dans la filière industrielle, parce que si on veut accélérer les énergies renouvelables, il va bien falloir qu'il y ait une filière industrielle qui soit créé pour le faire, et aujourd'hui nous sommes mis en difficulté et qui dit filière industrielle dit d'abord des savoir- faire et des compétences. Donc créer aussi aujourd'hui un certain nombre de compétences que nous n'avons pas par exemple si on parle sur le nucléaire, aujourd'hui, on voit bien que le fait sur les savoir-faire en matière de soudure nous mais en très grande difficulté donc quelle filière professionnelle nous créons puis les filières industrielles, après il y a le traitement des déchets, il y a la collecte il savoir le retraité, puis, à savoir le fabriquer et ce que vient de dire le président Gontard, il a tout à fait raison son Photowatt. Filiale 100 % EDF. Et EDF et le choix d'aller chercher du panneau chinois, donc là on a une contradiction complètement folle, hé oui, évidemment, sur le bilan carbone bah évidemment nos panneaux sont bien plus compétitif qu'ailleurs, mais aujourd'hui on est qu'aux prémices. D'un certain nombre de filières industrielles dans toutes les questions énergétiques, je reviendrai pas sur la vente de General Electric, vous voyez, on a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs en matière énergétique, et donc je vous le dis, Madame la Ministre, sur ce texte, il manque une base fondamentale sur quelle filière industrielle, vous allez vous appuyer pour accélérer le développement des énergies renouvelables, je vous remercie. pardon Monsieur Marchand. Oui, merci Monsieur le Président, en ce moment du débat, je pense qu'il faut aussi qu'on arrête un peu avec cette auto-flagellation permanente qu'on apprécie puisque on a quand même en France, c'est le PLF 2023 le démontrera, on a quand même quelques fleurons en matière de recherche aujourd'hui qui nous laisse augurer, j'ai envie de dire, de beaux jours je vais prendre pour exemple le CEA, l'institut Gustave Eiffel l'IFPEN énergies nouvelles qui sont aujourd'hui parmi les instituts qui ont les meilleurs classements en termes de dépôts de brevets dans le monde, ce qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai envie de dire que les pierres existe, il suffit de les assembler que bien évidemment, la nécessité de structurer la filière se fait sentir, mais que nous ne partons pas de rien. Merci bien, avant de passer au vote sur cet amendement va donner la parole à monsieur le rapporteur, puis Madame la Ministre. Oui, monsieur le Président, je voudrais simplement on va dire toute la confiance que j'ai, dans nos entreprises pour, à l'issue de la lecture de ce texte engagé vraiment le déploiement de de filière apporter quelques précisions sur la filière recyclage notamment pour Daniel sur les panneaux photovoltaïques, moi j'ai assisté en 2018 dans les Bouches du Rhône à l'inauguration d'une unité de démantèlement et de recyclage des panneaux photovoltaïques qui était conduite par un éco-organisme qui s'appelait à l'époque PV Cycle et qui s'appelle aujourd'hui, sereine, donc, la filière est organisé et à une une REP responsabilité élargie du producteur cette unité qui est gérée par Veolia permet de démanteler et de retraités jusqu'à 95 % du contenu du enfin du panneau en tant que telle et que par ailleurs, ça c'est une information pour mon collègue Guillaume Gontard mais qui, qui doit être parti particulièrement particulièrement voilà, je ne voyais pas informée, puisque la une nouvelle unité va se mettre en place, en Isère, dans son département, sur la même thématique et puis je voudrais citer également, plus récemment, une usine qui est une première du genre en Europe, hein, je, je, je vous lis, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui a répondu à un appel à projets de l'éco-organisme donc de recyclage, c'est en Gironde, ça s'appelle envie de The Aquitaine sélectionné dans le cadre d'un plan d'un appel d'offres, une usine qui permettra de de recycler, là encore 95 % des panneaux, ces 2 millions d'euros d'investissements, l'usine pourra traiter 4000 tonnes de panneaux par an avec 25 salariés en insertion, donc ça veut dire que cette filière de recyclage, elle existe, elle est mature, elle existe depuis 4 ans, il y a une râpe, donc, les opérateurs sont tenus de financer le démantèlement, la collecte le démantèlement et le recyclage des panneaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour pour la France, grâce à cette mise en place j'ai assisté en tant que président de du groupe d'étude d'économie circulaire, il y a 4 ans, et j'ai, j'ai pu le constater de mes propres yeux, voilà, c'était une précision que je vous apporter. Merci, monsieur le rapporteur, madame la ministre, avant de passer au vote. je vais être très rapide parce que, en fait, monsieur le rapporteur a a tout dit la Russie qui l'habilité des des panneaux photovoltaïques, c'est 95 % il y a un éco-organisme qui est en charge depuis 2015 et un certain nombre d'entreprises qui se développe, de ce fait, sur le territoire, avec plus de 15000 tonnes qui ont déjà été recyclés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je suis quand même rassuré, le Sénateur, Dantec sur le fait qu'on ne fait pas rien sur le nucléaire et sur l'organisation également du d'une filière puisque il y a des centrales qui seront démantèlement elle aussi avec des activités qui sont. Française et une vraie maîtrise et une vraie maîtrise française de cette filière tout n'a pas été fait, mais vous savez qu'il y a déjà eu des filière graphite des centrales graphite-gaz qui ont été démantelées et qui sont en cours de démantèlement et sur la question des des compétences et c'est une excellente question, elle se pose pour les énergies renouvelables, elle se pose pour le nucléaire, vous savez qu'il il y a des contrats stratégique de filière sur ces différentes différentes secteur industriel dans lequel nous avons des actions sur de formation et de compétences, je prends le nucléaire depuis 2 ans, nous avons des bourses spéciales pour orienter les élèves vers le nucléaire, nous prenons, nous formons du C. P jusqu'au bac plus cinq puisqu'on sait qu'on va avoir besoin de tous les métiers pour relancer un programme nucléaire et pour accompagner les grandes opérations de Karina De grand carénage, et cetera, donc sur ces métiers là on est dans une forme dans une phase de recrutement important et qui va dérouler dans les 20 années qui viennent, dernier point sur Photowatt je ne suis pas sûr que ce soit l'Alpha et une l'oméga de notre stratégie solaire, il se trouve que moi en 2010 au Fonds stratégique d'investissement, j'étais déjà sur le dossier de sauvetage de Photowatt, je l'ai croisée au Fonds stratégique d'investissement, j'ai 3 croisé quand j'étais à la Caisse des dépôts, j'ai croisé quand je suis devenu ministre de l'industrie, voilà, il y a peut être une une question plus profonde qu'on doit se poser, c'est comment on met en place des briques technologiques sur la filière solaire qui nous permettent d'avoir des panneaux photovoltaïques compétitif, compte tenu de ce qu'est le site France en terme de coût de l'énergie en terme de coût du foncier en terme de réglementation parce que, aujourd'hui, que ce soit tous tous les projets que nous on apporté, y compris de faire venir des investisseurs étrangers pour porter des se des projets je pense Arreckx Solar en en Moselle, hé bien, nous n'avons pas forcément les mêmes procédures procédures d'accueil, on va dire que d'autres, d'autres pays, je vous renvoie notamment à la lecture très intéressante du réduc une fashion acte qui vient d'être produit par le gouvernement américain et qui d'un point de vue de soutien financier déroule littéralement le tapis rouge, un certain nombre d'industriels des énergies renouvelables, vous savez que le commissaire breton s'est emparée de ce sujet là, mais je pense que ça doit nous poser au niveau européen et au niveau français, ça doit sauver de vraies interrogations sur ce qu'on fait dans notre stratégie, comment on accompagne les entreprises industrielles pour construire des sites au delà de la partie R&D innovation sur lequel on est effectivement assez solide. Bien, nous allons donc passer au vote sur l'amendement 536 présenté par Monsieur Houlgate. il est favorable à cet amendement. Qui est contre. Il est adopté. Alors maintenant, 3 amendements en discussion commune le 280 16 présenté par Monsieur Dantec. Merci monsieur le président, donc on a tous compris l'enjeu pour la France d'un développement rapide de sa production photovoltaïque à la nécessité d'une filière industrielle des filières de formation, on a déjà la filière de recyclage, donc le dispositif sur lequel on discute, a quand même une extrême faiblesse qui est finalement la la contrainte pour les exploitants qui ne voudraient pas équiper leur parking aujourd'hui, c'est extrêmement faible dans le texte, puisque peu prononcer. Et dans un limite de plafond de 10000 euros, on a parlé tout à l'heure des grands parkings des aéroports et moi j'étais pas obligatoirement totalement défavorable à l'amendement qui était proposé d'un peu de de souplesse sur ces très grands parkings et il est évident que vu les enjeux d'investissement 10000 euros pour un exploitant de très grands parkings pour ne rien faire et encore, c'est même pas sûr, il ne fera pas, s'il a pas envie de le faire, donc là je trouve qu'il y a une faiblesse très, très grande dans le dans le texte, donc on a repris la la calculette et on vous propose de déjà que la somme soit liée à la surface, c'est-à-dire qu'il ait une dix mille euros c'est pas la même chose pour un petit Parking ou un immense Parking et et que la la contrainte, soit à peu près, calculé sur le coût d'investissement, donc on vous propose 50 euros par place de Parking, ce qui correspond à peu près à 10 % du coût de l'investissement par an, donc ce qui est à peu près hein je pense dimensionné un niveau de contrainte acceptable qui n'est pas aberrant, donc voilà la la proposition, j'en profite, en 20 secondes pour dire à Madame la Ministre, de relire le dernier communiqué de l'ASN sur les graphite-gaz les caissons seront démontées en 2055 après qu'on ait un retour d'expérience du 1er caisson, donc on est quand même extrêmement loin du démontage des graphite-gaz. Ensuite, l'amendement 537 monsieur Houlgate. Oui, je pourrais dire qu'il a été défendu puisque c'est le principe justement de, de, de mettre une astreinte par mois de retard donc de de modifier le régime de sanctions.

nombres d'emplacements et non pas de surface au mètre carré pour définir son amendement, je suis favorable à cet amendement 296 qui opère plusieurs modifications bienvenues, ils ont laissé les sanctions plus progressive, on les rendant proportionnel au nombre d'emplacements, les sanctions seraient mensualisés sans augmenter le niveau global des amendes proposée par le projet de loi, par contre je suis défavorable à l'amendement 400 537 pardon qui reviendrait à multiplier par 10 le niveau des sanctions et à l'amendement 254 qui contribuerait même à multiplier par au moins 80 au niveau des sanctions donc restons-en là, au niveau des sanctions rendons rendons les progressive et proportionnelle. Madame la Ministre. Alors je, je, je vais donner un avis de sagesse parce que je pense que cet amendement pose différentes questions d'applicabilité mais j'en comprends l'enjeu, c'est de rendre cette obligation effective. Bien, donc nous allons soumettre l'amendement aux voix, enfin les trois amendements donc d'abord le 296 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, les 2 autres tombent, nous allons procéder au vote sur l'article 11 qui est favorable à l'article 11, ainsi amendé. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté. Donc, amendement après l'article onze l'amendement 451 présenté par Monsieur Gremillet.

à l'identique, c'est d'avoir une autorisation simplifié, allégé pour dans au niveau du code l'urbanisme, de manière à au renouvellement des installations photovoltaïques. Avis du rapporteur. Alors, je demanderai un avis de sagesse, une circulaire ou une instruction ministérielle ne pourrait-elle pas suffire pour distinguer clairement les renouvellements, procédant à des modifications substantielles et les renouvellement, procédant à des modifications de mon voilà je pose la question à la ministre et j'ai mis un avis de sagesse. Madame la Ministre. En fait, cet amendement, il est déjà satisfait monsieur le sénateur, puisque la partie législative du code de l'urbanisme prévoient à ces articles L. 421 1, renvoie à un décret en Conseil d'État pour arrêter la liste des Travaux sur constructions existantes devant être précédé d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable et les formalités sont d'ores et déjà prévues aux articles R 421 13 A R 421 17 1 du code de l'urbanisme, il n'est donc pas utile de prévoir un nouveau renvoi au décret spécifique pour les centrales solaires et puis mais vous le savez le cadre réglementaire actuel dispense d'autorisation d'urbanisme, les projets de renouvellement d'une centrale solaire dès lors que l'emprise au sol qui, n'étant pas l'emprise au sol, au delà d'un certain seuil, donc c'est une demande de retrait.

par les événements que nous avons subies en Gironde, les feux hors normes qui ont amené un certain nombre de questions et une des questions majeures, c'est comment constituer des zones d'appui et des pare-feu qui soit suffisamment efficace, mais comment créer des modèles économiques qui permettent, en créant ces zones d'appui et ses pare-feu, de pouvoir indemniser les propriétaires forestiers, or vous l'avez bien compris ses zones d'appuyer ses pare-feu doivent avoir aujourd'hui une dimension particulièrement importante pour être efficace, compte tenu de l'ampleur des feux que nous avons subi une des solutions, mais qui peut être une fausse bonne idée et de prévoir éventuellement l'installation de centrales photovoltaïques car il s'est avéré que celle qui a été bien entretenu, permettait de créer des zones d'appui efficace par rapport aux incendies, d'autres qui les témoins étaient parfois vecteur même de certains incendies il pouvait poser question, donc, en fait, cet amendement propose de mettre en place un rapport pour documenter véritablement le sujet et faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puisse prendre des décisions de manière éclairée sur l'intérêt ou non de créer des zones d'appui où des pare-feu sur lesquels nous pourrions installer des centrales photovoltaïques, d'où l'intérêt véritablement de créer ce rapport pour documenter l'ensemble des parties prenantes, voilà donc le but et l'objectif de cet amendement. Bien, merci, monsieur le rapporteur. J'ai répondu tout à l'heure sur un un autre amendement quasiment du même type, donc ce sera la même chose, même motif, même punition, entre guillemets, c'est un avis défavorable à cette demande de rapport ce sera traitée dans le cadre de la PPL dont dont j'ai parlé tout à l'heure. Madame la Ministre, également un avis défavorable. Bien don de double avis défavorable je soumets l'amendement on voit qui est pour.

La loi climat et résilience a introduit des nouvelles obligations sur le sujet, il y a un peu plus d'un an et afin de garantie la à garantir la stabilité logistique, il n'est pas souhaitable de modifier le quatre actuelle concernant les obligations de photovoltaïque sur toiture et par ailleurs la directive sur la performance énergétique des bâtiments est en cours de négociation. Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement, cet amendement de suppression revient évidemment sur une position qui a été prise par la commission donc je serai un avis défavorable. Madame la Ministre, ce sera un avis favorable. Donc un avis défavorable de la commission est favorable de Madame la mini-sur cet amendement de suppression de l'article qui est pour cet amendement.

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, notre amendement donc propose de rendre prioritaire : l'installation de procédés de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments commerciaux, industriels et de bureaux à construire subsidiairement uniquement lorsque de telles installations ne sont pas possible en raison de contraintes techniques de sécurité architectural ou patrimonial, un système de végétalisation pourrait être préféré. Merci Monsieur Salmon. d'accélérer la production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques, il faut vraiment aller dans ce sens-là et n'avoir une dérogation qui ne FIN& si il y a vraiment des contraintes trop importantes et qui ne permettent pas cette installation, donc je pense que vraiment il faut aller dans ce sens-là, merci.

Monsieur le Président, la miss, cet amendement vise à généraliser l'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable en toiture de toute nouvelle construction de bâtiment, l'usage d'habitation, il précise les conditions de la mise en oeuvre de cette obligation, les procédés de production d'énergie renouvelable en toiture devront couvrir une surface d'au moins égale à 30 % au moins égale à 20 mètres carrés dans le cas de maisons individuelles si l'implantation de ces dispositifs peut s'avérer complexe pour les constructions existantes hein marge de manoeuvre est importante en ce qui concerne les nouveaux bâtiments doivent être énergiquement performance sans quoi nous autoriserons des constructions obsolète. Je vais faire un parallèle à ce que moi j'avais pu mettre en place dans un lotissement libre de constructeurs et il y a quelques années, quand j'étais maire, j'avais imposée par exemple des cuves à eaux pluviales cubes sur chaque parcelle libre à l'acheteur de la parcelle d'en faire ce qu'il voulait et aujourd'hui ben tous les acquéreurs de ces parcelles ont effectivement utilisé ces ces réservoirs d'eau pluviale avant le rejet dans la nature parce qu'effectivement ça fait, vous allez faire des économies. Non négligeable : le 2ème amendement ben c'est le sable six cent c'est un amendement de repli, puisqu'il propose quand même de généraliser l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur toute nouvelle construction mais il renvoie au décret le soin de terminer les conditions d'application de cette obligation et le dernier amendement de mon collègue Bihac, il vise à supprimer toutes conditions restrictives, liées à la surface d'emprise au sol en ce qui concerne les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveau ou lourdement rénovée par des installations de production d'énergie solaire ou des systèmes végétalisée, comme a dit mon collègue précédent, bien que la commission et renforcer ses obligations en abaissant les seuils d'application à 250 mètres carrés, il convient d'aller plus vite et plus loin, en imposant à toute construction nouvelle de bâtiments non résidentiels, je vous remercie. Merci on examinera le le dernier après parce que d'abord les quatre en discussion commune, monsieur le rapporteur. nouveaux bâtiments non résidentiels j'ai toutefois une préférence pour le 540 qui fait entrer cette vie en vigueur cette obligation, au 1er janvier 2025 et laisse donc suffisamment de temps, porteurs de projets immobiliers pour s'adapter, avis favorable aux 540 et défavorable aux 209 sur le 603 rectifier cette génération bâtiments d'habitation de de l'obligation d'installation d'équipements ne me semble pas souhaitable cette obligation s'appliquerait à tous les bâtiments de plus de 20 mètres carrés cette obligation, c'est-à-dire beaucoup s'appliquerait à la promulgation de la loi, ce qui n'est pas réellement possible ou en tout cas, réaliste, je rappelle que notre commission déjà prévu de rendre les bâtiments neufs Solar Isabela c'est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables ah lactique, l'article 11 oct et que nous avons également adopté des dispositifs incitatifs par exemple l'éligibilité des panneaux photovoltaïques aux certificats d'économie d'énergie à l'article 11 7 Tia, ce sera donc un avis défavorable sur le 600 IV, là encore, l'obligation d'équipements, tous les bâtiments dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi pas réaliste, tout simplement, nous avons pris ou plutôt privilégier une logique progressive et en fait le calendrier que nous avons prévu 2027 et et à compter du 1er janvier 2028 pour le non résidentiel existant correspond en fait à celui proposé par la Commission européenne dans la directive performance énergétique des bâtiments, il y a une concordance avec ce que prévu, l'Europe, donc c'est un avis défavorable sur celui-ci. Madame la Ministre, sur ces quatre amendements. Alors sur le premier, un amendement, ça sera un avis défavorable, parce qu'au fond on pousse à retenir la solution photovoltaïque par rapport à la végétalisation, or la question de l'adaptation au changement climatique va quand même se poser de manière assez drastiques et donc laisser la possibilité entre les deux nous paraissait pas forcément infondées sur le 209 qui n'est pas si qui écrit de la même manière, c'est également un avis défavorable sur le 603 et le six cent vous avez déjà les l'impact de la réglementation et revint mais vous avez effectivement la directive efficacité des des bâtiments donc la direction qui est prise ici nous pourrait justifier un avis de sagesse, on risque de refaire bouger les lignes, avec l'adoption de la directive, efficacité énergétique des bâtiments, puisque vous le savez, nous avons adopté l'orientation globale en Conseil Énergie. Il y a 2 semaines, de mémoire et le texte final rentre en trilogue au niveau avec le Parlement européen et devrait être être adopté, si tout va bien d'ici la fin de l'année puisqu'on essaie de pousser pour avoir le maximum de texte pour faire que notre paquet climat-Hafid Fifty Five, soit le plus solide possible en entrée de de COP27 alors la COP27 c'est lundi, hein, mais il y a un certain nombre de textes qui sont en train d'être finalisé et en tout état de cause avec la présidence suédoise, qui prendra le relais, ça sera aussi un des textes qui sera finalisé, je suis entre sagesse pas. Que les sujets sont fondées et défavorable dans la mesure sur le premier des deux le 603 dans la mesure où il y a ce texte qui arrive et je pense que changer tout le temps la loi peut parfois être un peu compliqué. Bien, merci Monsieur Salmon. on voit après quelques années que ces ces toits végétalisés non quand même pas un apport très très conséquent, donc il faut effectivement privilégier les énergies renouvelables et, sinon, je demanderai à rectifier mon mon amendement sur le 540 s'il vous plaît, merci de rendre identiques. Bien, donc nous allons procéder au vote, donc d'abord sur le 540 rectifié et 209 puisque donc il vient d'être rectifié pour l'aligner sur le 540 avec un avis donc favorable de la commission sur le 540 et défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés ensuite le 603 rectifier. Dans la mesure où Madame le Ministre, pousse un peu, un avis de sagesse sur le 600 IV qui est plus généraliste et moins contraignant en matière de surface, je retire le 600 trois mais je maintiens le six cent. OK, donc je soumets au voile aussi son IV qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, donc le sur le 600 de qui a défendu tout à l'heure. Alors déjà présenté donc maintenu. Maintenu, monsieur le rapporteur, c'est un avis défavorable. Est également défavorable. Qui le présente monsieur Favreau. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, s'agit de de deux amendements qui suivent, qui sont de déclinaisons de l'obligation de superficie de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des constructions nouvelles, le 1er souhaite imposer une obligation sur la totalité de la toiture. remplace donc la formule actuelle du code de la construction et de l'habitation qui fixé cette obligation à 30 % le second qui paraît peut être plus raisonnables, fixe le taux minimum à 50 % quand on sait que l'orientation des peintures de de de chacune des toitures est quand même importante pour ce genre d'installation, c'est quelque chose à considérer et remplacerait donc le taux de 30 % qui est actuellement prévue par le taux de la construction et de l'habitation. Bien, merci, sur le 2ème amendement que vous avez présenté donc un amendement identique défendue par Monsieur Dantec. vous reconnaîtrez, comme toujours, la modération du groupe écologiste qui, malgré l'intérêt du premier amendement de notre collègue 100 % ça me semble quand même beaucoup et ça va poser quelques problèmes techniques, donc de manière raisonnable et on s'en excuse, on propose directement 50 %.

merci, ensuite un amendement monsieur Cabanel 606. Oui, cet amendement propose une un train vigueur du dispositif prévu par l'article 11 bis dans les 6 mois à compter de la promulgation de la loi. Et la main demain qui suit propose d'avancer de 2 ans, l'entrée en vigueur de l'obligation de couverture à l'énergie solaire, des bâtiments non résidentiels nouveau à dans le 1er janvier 2027 pour l'application d'une mesure qui pourrait rapidement train de vigueur et bénéficier aux usagers des bâtiments concernés ne nous semble pas raisonnable adhésion contexte de crise énergétique. Bien, merci, monsieur le rapporteur, sur ces six amendements en discussion commune. portée de 30 à 100 pour 100 de la surface de la couverture en énergie solaire des toitures des bâtiments neufs non résidentiels à compter du 1er juin mi-juillet 2023, c'est-à-dire demain, comme le propose l'amendement 169 me semble un peu excessif en revanche porter ce taux à 50 comme le proposent des amendements 170 299 et 539 me semble être une piste pertinent d'autant plus que ce nouveau taux ne serait applicable qu'à compter du 1er janvier 2025, nous laissons donc suffisamment de temps, porteurs de projets immobiliers pour respecter ce nouveau seuil c'est quand même assez récent, qui ne semble pas, a priori, poser difficultés techniques insurmontables insurmontable de passer de 30 à 50 on peut d'ailleurs imaginer que quand c'est possible, ont plutôt les ou les propriétaires ont plutôt intérêt à être à 60 70 ou 75 %, pour des raisons évidentes plutôt qu'à 30 ou 50, je rappelle d'ailleurs qu'il sera toujours possible de déroger à l'obligation de couverture des bâtiments non résidentiels neufs, du fait de contraintes techniques de sécurité architectural ou patrimonial si si cette obligation ne peut être réalisé dans des conditions économiquement acceptables, voilà et donc plus on monte le le taux, plus c'est intéressant sur le plan économique, donc c'est un avis défavorable sur le 169 et un avis favorable sur les 170 299 et 539 sur le 606 rectifié, je n'y suis pas favorable, 6 mois à compter de la promulgation de la loi, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très réaliste, enfin c'est pas du tout réaliste, notre commission a plutôt fait le choix de la progressivité en prévoyant d'assujettissement des nouveaux, des nouveaux bâtiments publics aux obligations de couverture en panneaux solaires dès le 1er janvier 2025, à cette même date, l'abaissement du seuil de l'obligation de couverture des nouveaux bureaux de 1000 à 500 mètres carrés l'abaissement du seuil de l'obligation de couverture des bâtiments non résidentiels nouveau de 500 à 250 dès le 1er janvier 2027 ce calendrier correspond là encore. Celui envisagé par la Commission européenne, ça nous évitera de revenir sur ce qu'aura intégré la directive et de modifier de nouveau on anticipe simplement avec ces dates et ces surfaces c'est donc un avis défavorable sur le 600 six même avis sur le six Donc, ça sera pour le 169 un avis défavorable, parce qu'effectivement 100 % % et vous l'avez dit vous-même, ne semble un objectif probablement inatteignable et qui peut poser un certain nombre de difficultés sur le 170 et le 299 je vais émettre un avis de sagesse dans l'incertitude de la fidélisation des négociations qui sont en cours au niveau européen, même si la direction qui est proposé paraît assez fondée, et par rapport aux enjeux du du texte sur le six six et le six

Bien, nous allons donc passer on voit monsieur Favreau, vous maintenez le le premier. Non, vous le retirer, donc je vais soumettre on voit directement les trois amendements identiques 170 299 et 539 avec un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient donc adopté, ça fait tomber le 600 six et je soumets aux voix le six Retiré OK. Donc nous passons aux amendements suivants : l'amendement 665 est un amendement de la commission monsieur Mandelli un amendement rédactionnel, monsieur le président, amendement rédaction. Lionel madame la Ministre. Alors comme il porte sur la rédaction de l'alinéa 6 du nouvel article onze bis les l'examen du projet de loi en commission avec lequel on n'était pas complètement d'accord, ça sera qu'un avis de sagesse. Donc un avis de sagesse du Gouvernement sur l'amendement de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je soumets aux voix, l'article 11 bis qui est pour cet article. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté, nous passons l'article 11 terre amendement de Madame avait, le 626. 626. Il est retiré, amendement 608 monsieur Corbizet. La Ministre, mes chers collègues, nous proposons par cet amendement de supprimer le critère lié au seuil de surface en matière d'obligations de couverture en dispositif de production d'énergie solaire, des bâtiments publics et commerciaux existants. Monsieur le rapporteur. réaliste donc je rappelle que ce serait d'ailleurs beaucoup plus contraignant, ce que propose la commission européenne, c'est-à-dire une obligation de couverture pour les bâtiments non résidentiels existants de 250 mètres carrés ou plus d'ici le 1er janvier 2028 c'est un qu'un un avis défavorable. Donc un double avis défavorable sur cet amendement, il est maintenu, il est retiré, pardon Monsieur Dantec, le 300. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement qui est attendu par une partie de la filière photovoltaïque française par des entreprises extrêmement performant notamment installé annonce je ne citerai pas de noms mais beaucoup savent ici de quelle entreprise je parle, c'est-à-dire on a vraiment une filière un un forte sur tout ce qui est photovoltaïque de façade avec des rôles en plus cumuler d'isolation des panneaux photovoltaïques qui laisse passer la lumière, donc il pleuvait sur les vitres, là il y a vraiment un savoir-faire français important donc cet amendement très simple permet juste en rajoutant ou de leurs façades d'autoriser c'est pas une obligation d'équipement hein, soyons bien clairs, c'est une autorisation d'équipements, je crois que là c'est un signal donné à cette filière française extrêmement performance en terme de recherche développement et qui a besoin de ces autorisations pour installer les panneaux. Monsieur le rapporteur. dans la définition, le bâtiment, dans son intégralité la toiture dont on parle souvent, mais aussi les les l'ensemble du bâtiment et et les façades, moi j'ai eu effectivement l'occasion de visiter en Loire-Atlantique, l'entreprise dont on parle à laquelle fait référence Ronan, c'est une entreprise qui aujourd'hui à des solutions qui sont mises en oeuvre, notamment en Allemagne et dans d'autres pays relativement peu en France parce qu'il y avait un un frein législatif, une entreprise qui investit quand je disais tout à l'heure que je faisais confiance aux entrepreneurs de notre pays et aux filières entreprise qui investit depuis 4 ans, 100 millions d'euros dans la recherche et le développement de ces nouveaux procédés photovoltaïque est installé à Chevrolet hier j'ai voilà, j'ai découvert dans le détail cette production pour préparer ce texte avec d'autres visites dans d'autres entreprises de secteur et collectivités, donc c'est un un avis très favorable pour que l'ensemble des solutions pour éviter de consommer des espaces au sol et sur les toits, on peut voilà en mettent beaucoup sur la voiture, mais on peut aussi en mettre énormément sur les façades, donc c'est un avis plus que favorable, mon cher collègue. Madame la Ministre. C'est un avis défavorable, car la loi climat et résilience a introduit dans son article 101 de nouvelles obligations de couverture de toiture, il y a un peu plus d'un an, les textes d'application sont en cours de finalisation, l'article 11 terre nuit à la lisibilité du dispositif existant, car il est redondant en partie avec les dispositions de la loi climat et résilience est incompatible, notamment s'agissant de la végétalisation des des c'est pourquoi la le gouvernement avait émis un avis défavorable sur l'amendement ayant introduit cet article onze terre, par ailleurs, la directive performance énergétique des bâtiments, reprenant la mesure du plan are You, de la Commission européenne relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments est en cours de négociation, donc on risque de devoir devoir avoir des des alignements, la priorité est aujourd'hui donné en France comme au niveau européen en développement des énergies renouvelables et de la végétalisation en toiture mélangé ses obligations, avec des dispositions relatives aux façades et de nature à nuire au message et donc nous souhaitables, à ce stade.

de recherche et d'implication française qui vient en même temps de de récupérer une entreprise américaine pour développer la production française aux États-Unis si on monte un un signal en disant : écoutez on vous complique les choses et pour le moment, vous ne pouvez pas aller sur les façades et aux photovoltaïque, je crois qu'on fait on on est en train de les freiner et de et de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer aux États-Unis complètement aux États-Unis, après ils viendront à partir des États-Unis développer leur leur production en France.

dans les décrets d'application et je ne vois pas pourquoi au niveau européen, ça, ça rendrait les choses plus compliquées, tellement il est évident aujourd'hui, ça a été dit l'Allemagne il va rapidement en quoi ça serait plus compliqué de rajouter les, les, les façades dans dans le décret global, donc je crois qu'il faut effectivement voté cet amendement et on compte sur l'administration française pour faire en sorte que les décrets intègre les façades. Bien, donc nous allons voter cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, l'amendement 300 hein Non, mais il vous a pas échappé qu'il m'arrive de voter vos amendements aussi hein, sauf, sauf quand ils vont trop loin en terme d'objectifs écolo rapide donc cet amendement en fait fait écho à l'amendement précédent sur les parkings, que nous avons d'ailleurs tous voter et je remercie le rapporteur Mandelli, non seulement pour les avis favorable et pour tout le travail qu'il qu'il développe depuis plusieurs semaines, on a le même problème en fait sur les toitures, qu'on avait sur les parkings avec une une pénalité s'il n'y a pas équipements qui est trop faible dix mille euros c'est vraiment pas beaucoup par rapport y compris avec les les contraintes à 10000 euros il y a des propriétaires qui qui n'iront pas, donc là on n'a pas réussi à faire le même calcul parce qu'on n'a pas les mêmes différences de surface entre les toi il y a pas des 3 2000 mètres et des toits de de 50 hectares, donc on a préféré remettre une une c'est discutable la logique aurait été de mettre probablement un pourcentage mais le calcul était plus compliqué, donc 10000 en tout cas c'est très peu, donc on l'a monté à 25000 ce qui reste aussi raisonnables. Oui, c'était le trois cent de là, je peux donner de réponse. Oui, oui, excusez-moi, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mais j'ai, j'étais encore tout à la joie de l'amendement précédent adopté

ben il va être défendu, hein, pour gagner du temps et je m'excuse. Alors, monsieur le rapporteur sur le 300 hein. Oui, monsieur le Président, l'euphorie de notre collègue va vite retomber, puisque je vais donner un avis défavorable à retrouver un équilibre dans un souci de cohérence avec ce que nous avons monté avec le dispositif existant en matière de couverture, nous avons fait le choix de laisser l'autorité compétente, définir les situations dans lesquelles il pourra être dérogé à l'obligation de couverture des bâtiments, donc c'est un avis défavorable. Défavorable. Donc un double avis défavorable, il est retiré le 607 monsieur Corbizet.

la réglementation européenne sur les 250 mètres carrés donc là effectivement ben tout simplement se présent amendement propose d'avancer de 4 ans, l'application des obligations d'installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics et commerciaux existants,

Défavorable également. Donc double avis défavorable Monsieur Gontard. des bâtiments, des bâtiments existants sur quelque chose qui n'est pas du goût qui est qui pour le coup, réglementaire et qui est pas de législatif mais sur les seuils de tarifs d'achat puisque ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces seuils de 0 à 36 kilowatts crête à 36 à 100 et de 100 à 500 etc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le le lissage de ces seuils, puisque sur l'équipement de de toiture, ces seuils souvent mène à faire en sorte que on équipe à la totalité de la toiture pour des questions de rentabilité liée justement au tarif d'achat et ce qui est pour le coup très dommageable alors qu'on pourrait utiliser l'entièreté de la toiture, donc je pense qu'il y a une une réflexion à avoir justement sur ces, sur ces seuils et le lissage de ces seuils, pour permettre en tout cas, qui a même un bonus pour quelqu'un qui utilise la totalité de la toiture. Merci. Bien, merci donc à un double avis défavorable mais l'amendement est retiré, donc le six de qui a déjà été présenté par Monsieur Dantec. ça, ça ne vous avez pas échappé qu'il a déjà été défendu.

Les comptes. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, donc je vais soumettre au au votre, l'article 11 terre qui est pour cet article.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que l'accélération de la production d'énergies renouvelables se confronte à la nécessaire préservation des Terres agricoles naturelles et forestières, il est primordial de facilité de développement des énergies renouvelables, sur les zones déjà artificialiser le potentiel énergétique et grand selon l'Ademe, nous pourrions installer 53 gigawatts du photovoltaïque sur des zones déjà artificialiser et 7 gigawatts à très court terme, comment pouvons-nous ignorer cette réalité alors que notre objectif commun est d'accélérer le développement des énergies renouvelables au delà des parkings, des bâtiments commerciaux nous devons encourager l'installation d'énergies renouvelables notamment photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments ainsi l'amendement que je vous propose adopter vise à soumettre les permis de construire et les déclarations préalables à la réalisation d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable la réalisation d'une étude de faisabilité permettra d'anticiper la viabilité et les implications économiques org a organisationnel d'un projet d'installation d'énergies renouvelables, elle sera un outil précieux pour les propriétaires, loin d'être Kirsty Steve, l'étude de faisabilité vise à inciter les acteurs privés et publics, en révélant le potentiel énergétique de leurs bâtiments. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, soumettre les permis de construire et des déclarations Perrin là-bas la réédition d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement d'énergies renouvelables, me semble, hein, j'en ai acquis la certitude, le parc Armand lourd tant pour les personnes sur la distance et les permis de construire et ses déclarations préalables que pour les services instructeurs de plus, je suis pas certain que cela contribuerait concrètement accélérer le déploiement d'énergies solaires en toiture par exemple ce que rien n'assure en effet que les projets soient déployés après la réalisation de l'étude. Donc pour moi c'est un un avis défavorable je fais confiance là encore aux entreprises, aux particuliers à tous aux architectes qui pourront, dans leur démarche aux maîtres d'Oeuvres, proposer des solutions de ce type, donc c'est un avis défavorable à ce stade, on ne peut pas obliger tout le monde va faire une étude préalable. madame la Ministre avis défavorable également. Donc double avis défavorable je soumets l'amendement voix. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté amendements suivants monsieur Cabanel le 458. Si Monsieur le Président, nos concitoyens ne sont pas toujours au fait de l'existence d'un ensemble de dispositif de soutien public accompagnant l'installation d'équipements de production d'énergie solaire et les possibilités qui s'offrent à eux pour les intégrer dans leur construction le présent amendement vise à inciter les demandeurs d'un permis de construire ou d'aménager à la réalité réévaluation pardon de leur projet, pour étudier la faisabilité de ces options et pour cela, il est proposé de les orienter vers le service de la performance énergétique comme Pétain lors du dépôt de leur demande. Sur le rapporteur, c'est à peu près le même commentaire que sur l'amendement précédent et ce sera un avis défavorable. Défavorable. Donc un double avis défavorable je soumets l'amendement, on voit qu'il est retiré. Bon tirer. Amendements suivants Monsieur Salmon, le 210. Merci monsieur le président, madame la ministre, on l'a bien entendu, hier, de la part de certains collègues le monde rural, estime qu'il fait beaucoup pour les énergies renouvelables, il faut surtout pas opposer les territoires mais bien parler de complémentarité, mais je pense que la ville, le monde urbain doit aussi optimiser son potentiel et donc cet amendement va dans ce sens parce que les bâtiments collectifs d'habitations sont un gisement très importants de production énergétique notamment photovoltaïque en raison des surfaces importantes que représente non seulement les toits mais en ville, surtout les façades, on en a parlé tout à l'heure avec l'amendement de mon collègue Dantec afin d'accélérer le développement de ces énergies renouvelables, les règles relatives à l'installation d'ouvrages de production d'énergie dans les copropriétés doit être facilitée donc cet amendement propose de simplifier, afin que les travaux relatifs à l'installation des dispositifs de production d'énergie puissent être pris à la majorité simple des copropriétaires parce qu'aujourd'hui il faut une majorité qualifiée qui est beaucoup plus difficile à atteindre, tout ceci au même titre que les travaux d'acceptabilité d'accessibilité PMR et aussi les travaux d'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, donc on voudrait les mêmes règles pour les installations photovoltaïques. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, nous avions eu à peu près le même genre de de réflexion d'interrogations au moment de la loi d'orientation des mobilités pour l'installation des bornes de recharge sur sur sur les parkings avec donc de, de GoPro, cet assouplissement des règles que vous souhaitez me semble être une piste intéressante pour accélérer le déploiement dans les immeubles résidentiels, toutefois je j'aimerais connaître l'avis du gouvernement, parce que, à ce stade, voilà, j'ai un peu de doute malgré tout. Madame la Ministre. des copropriétaires à ce type de décision à la majorité simple, telle que vous le proposez peut conduire à avoir une décision qui est prise à une très faible majorité de de copropriétaires est porté à une atteinte disproportionnée aux droits des copropriétaires sur les parties communes avec ensuite des difficultés dans la mise en oeuvre de la décision et donc il vaut mieux s'agissant d'opérations qui ont quand même un impact assez important sur la copropriété c'est pas tout à fait la même chose que mettre une borne de recharge et qui suppose des financements importants s'assurer d'une volonté réellement partagé avant l'engagement de ce type d'opération. Merci madame Prima, beaucoup d'immeubles logements sociaux en copropriété dans lequel le bailleur social est majoritaire, mais il y a des copropriétaires et qui sont des copropriétaires modestes issu du monde ouvrier automobile et qui ont acheté peuchère, ces appartements, dans des conditions il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils n'ont pas les moyens de faire ça, sauf à être accompagnés par des dispositifs d'État très important, ils n'ont pas les moyens de faire ça donc je, je, je comprends l'esprit d'accélération, en revanche, vraiment il faut être très très prudent sur la règle de copropriété, notamment sur les copropriétaires très modeste. Oui, je pense qu'on a, on a 2 questions différentes, c'est très très difficile aujourd'hui d'avoir des décisions de copropriété au-delà la majorité simple, parce que les gens ne viennent pas, donc, donc, si, si on cherche une un autre type de majorité, rien ne se fera donc c'est le sens de l'amendement de de Daniel Salmon, mais j'entends tout à fait ce que vient de dire Sophie Primas et là je pense qu'on est sur une autre question et qui est d'une des questions centrales qu'on ne traitera pas dans cette loi, malheureusement, qui est la question du financement là typiquement, on doit être sûr du tiers investissement : il ne faut pas que ça, ça soit un investissement évidemment des des propriétaires mais est-ce que l'amendement Daniel Salmon hein pèse le tiers investissement je je ne crois pas, mais en tout cas je crois qu'on doit tous conscients que si, en plus de tout ce qu'on est en train de faire pour faciliter, effectivement, l'équipement photovoltaïque des parkings, des toitures et de plein d'endroits où on n'a pas du tiers investissement et probablement comme ça se passe aujourd'hui en Allemagne qui avance extrêmement vite sur le renouvelable, même si des fois, on entend des choses inverse en Allemagne, c'est l'équivalent de la Caisse des dépôts qui aujourd'hui multiplie les outils financiers pour accélérer, on a besoin de la même chose en France, donc moi j'entends tout à fait ce qu'elle dit Sophie Primas mais c'est pas la même question : si on sort de la majorité simple, on ne fera rien.

voir dans quel contexte on est aujourd'hui, et bien entendu, je ne veux pas prendre ce qu'a dit mon collègue Dantec, mais effectivement les populations à revenus modestes, il faut qu'il y ait des tirs enfin une financeurs, sinon on va pas y arriver mais il faut s'inscrire aussi dans dans la dynamique de l'accélération et le fait que l'énergie devient de plus en plus coûteuse et ces investissements sont des investissements qui vont apporter une rentabilité a plutôt court terme. Cette question là, nous l'avons évoqué avec le président de la commission et certains des rapporteurs de groupes politiques, lors d'une réunion au ministère effectivement quand on sait que la prévenue ne rénovent ne fonctionne pas bien les, on sait que les classes moyennes pour effectivement investir dans du photovoltaïque ou d'une forme durable il y aurait plus de développement,

et lors du réunion à mystère, on avait évoqué la possibilité et ça ne sera pas dans cette loi-là mais peut-être dans une loi de finances, que les gens qui freine l'investissement sur les économies d'énergie et donc baisser leurs leurs dépenses de fonctionnement puisqu'ils auraient dû l'autoconsommation, si on pouvait effectivement dans une loi de finances, imaginer que ce qu'il ferait un emprunt pour faire des économies d'énergie, ce ce, ce taux d'emprunt pourrait ne peut être ne pas intégrer le l'endettement des à se rajouter à l'endettement de de l'accession à la propriété, donc il y a peut-être une solution à trouver pour effectivement de d'accélérer le développement des de l'autoconsommation avec ce qui aurait les moyens de le faire. Bien, merci, donc on a un avis défavorable du gouvernement et, finalement, de la commission qui est la vie. C'est très clairement sur cette question parce que il y a des éléments qui ont été apportées, moi je, je pense que si on a ouvert la possibilité, dans, dans, dans le texte à la fois de faire de consommation et en particulier avec des tiers investisseur je pense que dans le cas précis, si effectivement il y a un tiers investisseur qui arrive, qui propose l'autoconsommation et que ça ne remet pas en question, les propriétaires ou la co-prod aura tout le loisir avec ce qu'on a déjà mis dans le texte de faire sans avoir besoin de modifier les règles de vote l'assemblée parce que le droit s'imposera, ils pourront décider si ça leur coûte rien évidemment de, de, de prendre, donc il y a pas de frein à la mise en place avec des petits investisseurs dans le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui sur ce type d'opération, donc il y a aucune raison effectivement où maintenant et cure de à la fois de la vie de la ministre et ce que j'ai entendu donc, moi, à mon avis, de sagesse va plutôt, j'avais demandé l'avis du gouvernement, avis de sagesse, mais ce sera plutôt un avis défavorable. Bien, donc un un double avis défavorable je soumets l'amendement voix qui est pour.

Alors Monsieur. Ah pardon, excusez-moi, allez-y, l'amendement 538. Oui, monsieur le président, donc, dans le cadre de ses travaux, la commission a introduit la possibilité de déroger aux interdictions prescrite dans les règlements des plans de prévention des risques inondation à l'époque des PPRI, pour le déploiement d'installations de production d'énergie solaire, or nous n'avons pas d'étude d'impact sur la maîtrise des risques que pourraient présenter une implantation de projets photovoltaïques au Sol en zone inondable aussi notre amendement de suppression est un amendement d'appel pour recueillir l'avis du gouvernement sur ce sujet. Merci de la commission. Oui, un avis défavorable, cet apport pragmatique qui a été introduit en commission permettra de libérer des espaces à faibles enjeux fonciers pour le déploiement des énergies renouvelables, dispositif est plutôt bien encadré avec un rôle pilote du préfet

Donc un avis favorable de la de madame la ministre, et un avis défavorable de la commission. Donc je soumets oui sur l'eau. Oui, je crois qu'il faut argumenter ce cette proposition le le risque inondation, aujourd'hui il est réel, il existe d'une manière c'est un peu l'épée de Damoclès pour les populations qui vivent dans ces zones là il y a des crues décennales, centennales 5 centennale et aujourd'hui les documents d'urbanisme font apparaître que, à défaut de risques avérés, il y a des modélisations qui permettent par exemple de contenir l'urbanisation et les modifications qui sont apportées au. au. Plans locaux d'urbanisme, donc il y a un risque réel, y compris pour les gens qui ont déjà un pavillon pour lesquels on leur dit, par exemple, de construire une véranda, ça n'est pas possible puisqu'ils sont en zone PPRI et donc ce risque inondation avec le réchauffement climatique il perturbera de plus en plus les secteurs qui sont impactés et c'est la raison pour laquelle toute modification de l'urbanisme, y compris, y compris implanter des panneaux photovoltaïques ou quelque chose qui, qui qui ne présentent pas apparemment un danger ça nous paraît quelque chose qu'il faut contenir et en tout cas c'est une démarche de protection des populations et de, de, de précaution à l'égard de, de, d'une urbanisation sauvage, même si on comprend parfaitement qu'il faut accélérer le rythme de déploiement des énergies renouvelables. La présidente Sophie Primas. Oui, merci Monsieur le Président, moi je vais soutenir la position de la commission du développement durable sur ces zones en PPRI, ce sont des zones dont on ne peut rien faire, pas grand chose en tout cas et dans lequel il me semble qu'il y a des nouvelles technologies style ombrière sur des pieds alors j'y connais rien, excusez-moi, mais enfin il me semble qu'on peut mettre les panneaux photovoltaïques un peu en hauteur en regardant le niveau des crues dans les dernières années, peut-être en le multipliant par 2 en se disant que ça va être pire, dans les années prochaines, mais il me semble que technologiquement on peut utiliser ces espaces là pour installer précisément sur ce terrain dans lequel on ne peut pas faire d'urbanisation, et cetera des des champs de photovoltaïque, il me semble, en tout cas que c'est plus raisonnable de soutenir la la la dérogation qui est prévu par la commission. Monsieur Dantec. Oui, je fais moi tout à fait dans le sens de de Sophie Primas c'est on, on, il y a des zones à risque, mais on ne va pas les les gelées, sauf si elles ont un grand intérêt de reconquête de la biodiversité, la part des choses, donc au contraire, il faut, il faut savoir utiliser ces zones sur des risques qui ne sont pas des risques sans trop pour l'activité humaine donc donc je je suis complètement comme Sophie Primas comme la commission je je ne vois pas l'intérêt de cette restriction. Bien, donc nous allons soumettre l'amendement au au vote qui est favorable à cet amendement. Qui s'abstient, Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Ah, ensuite un amendement présenté par monsieur Mandelli au nom de la commission, un amendement rédactionnel, monsieur le président. Amendement rédactionnel madame la Ministre, pas de remarques sur cet amendement, l'amendement 666. Favorable ou défavorable à pardon défavorable, excusez-moi, donc je soumets cet amendement rédactionnel de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, je soumets aux voix, l'article 11 quater, qui est pour cet article. Qui est contre qui s'abstient il être adopté. Nous passons l'article 11 qui inquiète avec 2 amendements identiques de suppression. Le premier, le 197.

cette mesure ne nous paraît pas justifiée dans la mesure où les gains en termes de production d'énergie très très faible, alors qu'elle aurait des conséquences très forte sur le Cadre de vie et l'attractivité touristique de certains territoires, je rappelle que l'avis conforme des ABF ne concerne qu'une partie restreinte du territoire national et que le taux de refus de ces projets dépasse à peine les 10 à cela s'ajoute le fait qu'un travail a été engagée par le ministère de la culture et le ministère de la transition énergétique pour faciliter le déploiement de panneaux photovoltaïques en espace protégé qui nous paraît faire perdre à l'article 11 qu'inquiète une grande partie de son objet en effet les 2 ministères devraient avant la fin de l'année, publié une instruction destinée aux services déconcentrés en charge du Patrimoine cette instruction définira des lignes directrices à destination des ABF sur la manière dont ils doivent traiter les demandes d'installation de panneaux photovoltaïques, l'objectif serait notamment d'autoriser le déploiement de telles installations dans tous les secteurs des espaces protégés à faible enjeu patrimonial comme les zones commerciales, industrielles, les parkings des zones pavillonnaires et même les bâtiments dont la construction est postérieure à 1948 dès lors qu'il n'y a pas de problème de cadrage paysager dans ces conditions, l'installation de panneaux photovoltaïques dans ces espaces ne devrait plus vraiment soulever de difficultés, mais notre Patrimoine restera protégée grâce au contrôle opéré par la BF. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en fait, cet amendement, hé bien est identique à celui que vient défendent la rapporteure pour avis Madame Garnier je ne vais pas refaire mon couplet sur les ABF nous en avait des, nous en avons déjà discuté hier simplement je voudrais quand même au dire 3 choses : la première c'est, contrairement aux idées reçues, il faut quand même que vous sachiez que les avis des ABF ne ralentissent pas toujours les projets et signifierait en tout cas ne ralentissent pas toujours toujours significativement les décisions et encore moins le déroulement des différentes opérations d'aménagement, je trouve que c'est toujours intéressant, mais je sais, je vois, je vois la prison de la cuisson des affaires économiques, le dire, mais c'est intéressant toujours sont des garde-fous essentiel et et les avoir autour de la table, c'est important, comme on vient de le rappeler, comme vient n'a rappelé la rapporteure, seuls 10 à 10 pour 100 des avis concerne les projets d'installations photovoltaïques qui aboutissent aujourd'hui à des refus de l'opération projetée, il ne semble donc je voudrais vous rappeler enfin que la création des sites patrimoniaux remarquables est récente : elle remonte à la loi du 7 juillet 2016 qui a permis de regrouper sous une seule appellation les anciens secteurs sauvegardés que nous connaissons les aides PPA les ah vap'et surtout, et ça c'est important d'unifier le régime de protection et d'autorisation lorsque des travaux, ils sont envisagées, donc je pense qu'ici il ne s'agit pas encore d'entraver l'ensemble des projets d'installations photovoltaïques, mais simplement d'entourer des garants de garantie, ceux qui sont susceptibles d'affecter le Patrimoine de nos concitoyens. Bien avis de la commission sur ces deux amendements de suppression. Oui, monsieur le président, cet article est un introduit en commission, via un amendement sur lequel j'avais donné un avis de sagesse, pourquoi un avis de sagesse parce que évidemment j'étais très partagés sur cette question quand j'entends la porteur Laurence Garnier je comprends ses préoccupations, je partage en grande partie en matière de protection mise en valeur du Patrimoine comme chacun d'entre nous, on l'a d'ailleurs évoqué hier quand on a aussi parlé des ABF, de l'autre, en tant qu'élus locaux en tant qu'acteur, des territoires, nous savons que les ABF bien sûr ont un pouvoir bloquant qui est parfois déraisonnables et surtout des interprétations qui, d'un département à l'autre, d'un secteur à l'autre sont très très variable, un changement d'ABF peut donner un changement d'avis et et c'est très inégal d'un département à l'autre, ce qui empêche évidemment de développer des projets qui sont pourtant utile et porté par les papes population locale et les élus, c'est ce qui a expliqué les nombreux amendements déposés en commission à ce sujet et le vote de la commission pour leur adoption. Depuis le vote en commission, on a eu évidemment l'occasion d'échanger avec Laurence Garnier avec beaucoup d'autres, le fait d'avoir eu confirmation qu'un travail était engagé entre les 2 ministères pour tenter d'harmoniser, de prendre en compte ce développement des énergies renouvelables, éventuellement d'autres sujets m'a fait évoluer et je donnerai donc un avis favorable aux amendements de suppression 197 et 519 mais je souhaite que la ministre nous confirme que ce travail a bien été engagée entre les 2 ministères et qu'il aboutira à priori, c'est ce qu'on m'a dit correspond en en début d'année à l'élaboration d'une charte pour harmoniser les positions et prendre en compte les souhaits des élus locaux. Madame la Ministre. sur le terrain des situations où j'ai du mal à expliciter les positions qui sont prises et, effectivement, c'est encore plus difficile pour les positions changent d'une fois sur l'autre ou d'un dossier à l'autre, donc nous avons entamé avec le ministère de la culture, un travail méthodologique, il s'agit d'avoir un guide, mais encore faut-il que que ce guide soit complètement je dirais partagé qui est aussi à à un partage de bonnes pratiques entre les APF et probablement des lignes ferme sur ce qui relève de la protection du Patrimoine et ce qui relève peut-être de l'appréciation un peu plus personnelle et de, de manière à rester sur la protection du Patrimoine, donc le travail est entamé, il est encore très préliminaires, hein, je veux pas vendre du rêve aujourd'hui, mais je pense qu'il faut donner sa chance à ce travail, il est important que sur le territoire, on est une homogénéité de la de la mise en oeuvre de notre politique de protection du du Patrimoine, et moi je, je ferais un avis favorable à cet amendement parce que je souhaite que ce travail se déroule dans les meilleures conditions. La présidente Sophie Primas. mais nous savons tous ici, non, je n'ai rien contre les ABF, au contraire, je trouve que quand on travaille bien avec elle, c'est une opportunité de bien faire les choses donc je, je n'ai rien contre Isabelle j'ai j'ai contre le fonctionnement parfois solitaire

il faudra qu'on regarde comment ce guide pourra être opposable ou pas. Parce que c'est un sujet si c'est un guide pour un guide et que derrière il y a pas de pause, comment on pourra l'utiliser mais je voudrais dire quand même, on ne faut pas se cacher la face, il y a quand même des projets, on en a tous dans nos territoires et je pense, quelles que soient les bancs et quelle que soit la commission chers collègues dans laquelle on siège où on a des projets qui sont bloqués ou qui sont même arrêter définitivement et qui sont pas faisable, alors que franchement, on peut se poser la question du pourquoi donc voilà, je trouve que l'amélioration les souhaitable, elle est, elle est vraiment souhaitable parce qu'on a besoin des ABF pour protéger notre Pratt Rimons mais il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'on puisse un peu à avoir des explications et un travail en commun avec les ABF, je reconnais qu'en fonction des ABF c'est faisable ou pas, c'est bien ça justement qui est regrettable. les antennes de téléphonie mobile, il se trouve qu'avec ma collègue Anne, nous avions fait, nous avons fait récemment un rapport sur l'état des édifices religieux et il nous est remonté que dans de nombreuses combines aujourd'hui les clochers d'église se retrouver avec des antennes de téléphonie mobile, c'est la conséquence immédiate du du travail de sape que vous avez fait sur l'avis conforme des ABF, donc on peut continuer, et a ajouté maintenant des panneaux photovoltaïques sur les églises, ce que ce que j'aimerais vous rappeler parce que c'est tout à fait essentiel c'est que la France est la première destination touristique mondiale, le Patrimoine, c'est un investissement, c'est pas une charge, c'est un investissement, c'est ce qui nous permet d'accueillir tous les ans des touristes de plus en plus nombreux, donc il faut travailler sur sur sur cet aspect qui est tout à fait essentiel ensuite, madame la ministre, vous êtes au banc du gouvernement, c'est-à-dire que vous défendez aussi les intérêts du ministère de la culture, je suis surpris de vous entendre attaquer les positions divergentes des avis des des oui, mais c'est un constat qui vont, qui va dans le sens des élus quand ils attaquent des ABF, je crois que c'est pas le rôle du gouvernement autre point le ministère de la culture et un train de préparer des des instructions nationales très précises qui correspondent tout à fait ce que demande la la présidente Prima de ce que j'ai compris le travail du côté du ministère de la culture et et achevée et achevé Madame la Ministre, il a achevé non. Il est pas achevé parce que vous le bloquer non parce que vous le bloquer, c'est ce que nous a dit : le ministère de la culture aujourd'hui le travail a rendu c'est de votre côté, qui a un problème, donc vous voyez, vous voyez, donc là il faut il faut retourner, donc c'est votre travail, qui est en cours, merci monsieur le président. Merci monsieur le président, chers collègues, j'avais prévu d'intervenir pour défendre cet amendement mais finalement je je viens au secours de la victoire, d'après ce que ce que j'ai compris c'est c'est c'est assez agréable également juste un mot quand même l'objectif de la loi, c'est de développer les énergies renouvelables, l'objectif de cet article, c'est, c'est c'est de revenir sur le mode de fonctionnement des architectes des Bâtiments de France on l'a dit l'enjeu en terme de développement d'énergies renouvelables dans les périmètres classés dans dans les proportions de de de co-visibilité qui aboutirait sur un un avis défavorable, il est minime par rapport à ce qu'on vient d'étudier sur les les ombres hier sur les toitures des bâtiments existants sur les bâtiments futur et cetera, je pense que la filière chinoise a largement assez à faire

combien de bâtiments qu'on a réalisé depuis 20 ans, parfaitement étanche isolée par l'extérieur et seront encore visitables dans un siècle ou dans 2 siècles, combien plus aucun préservons au moins ce que nos prédécesseurs ont fait, c'est notre bien commun, c'est un Patrimoine qu'on qu'on qu'on se doit de préserver, c'est une richesse de notre pays et donc c'est un enjeu qui est majeur, l'enjeu de de des des villages médiévaux de de des sites patrimoniaux avec les panneaux photovoltaïques pour lequel on est favorable, il y a d'autres endroits pour les mettre mais comme comme comme par l'isolation par l'extérieur, on a aussi ce ce genre de difficultés où les maires se retrouvent en difficulté face à des pétitionnaires, l'appui de la BF et l'avis éclairé de la BF être important, moi aussi, on a souvent été en en confrontation avec la BFC c'est normal on on échange, néanmoins, on est dans une situation où il a un rôle important, celle-ci en en fait partie. Merci, cher collègue, il y a beaucoup d'inscrits en Monsieur Pointereau. Monsieur Pointereau. Bilan : Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est vrai qu'il y a parfois des différences d'appréciation d'un département à l'autre, vis-à-vis des bâtiments de France, et ça pose des problèmes on arrête tes projets pendant un certain nombre d'années avant de d'aboutir, mais là pour le coup, c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude des maires qui ont parfois des petites villes de caractère ou des patrimoines leur, dans leur commune et qui ont peur de voir fleurir des toitures de photovoltaïque à proximité et ça, ça risque de poser des problèmes de, de Patrimoine, parce qu'on a quand même un Patrimoine en France important et je pense que pour le coup, moi je soutiendrai évidemment le l'amendement de notre collègue Laurence Garnier qui va permettre de de protéger parce qu'à un avis simple ça peut parfois un petit peu déroger, et il y a déjà une d'ailleurs un comité de concertation au niveau des départements pour déroger parfois au aux avis des des bâtiments de France avec la la préfecture, donc ça permet déjà d'avancer mais là si a la un avis simple et il y a eu une discussion déjà dans la, je crois que c'est au niveau de la loi élan où on avait une une discussion importante vis-à-vis des des architectes des Bâtiments de France, où on voyait bien que les choses allaient parfois et on a, on avait finalement retenu cette volonté de concertation avec les Bâtiments de France pour avancer par, par contre, par rapport à ce que disait tout à l'heure notre collègue vous alias les les antennes au niveau des clochers, j'en ai pas vu beaucoup, ils sont allés à l'intérieur des clochers, souvent ils sont posés à l'intérieur, donc là ça pose pas forcément de problème mais là pour le coup, le le photovoltaïque sur des petites cités de caractère, ça serait quand même vraiment dommageable. Merci Monsieur Dantec. Oui on on est sur un débat avec plus, plusieurs questions assez différentes : la première, je crois c'est que effectivement le fonctionnement actuel donne un rôle à des individus sans que les les cadres soient clairement fixé, c'est ça la première clairement des injonctions contradictoires et que ce ce système effectivement, c'est ce qu'a dit Sophie Primas est extrêmement problématique dans dans beaucoup d'endroits et donc effectivement il faudrait il y a à voir des cadres de l'État, mais je crois que ça a été dit les uns et les autres ne défendent pas exactement les mêmes priorités, donc moi je pense que c'est en rester à la logique de la vie conforme, faute de mieux, c'est c'est de plus en plus fragilisé le système même des ABF et qu'il faudrait effectivement des cadres clair écrit entre les ministères, validé par le gouvernement et qui s'applique à tous, le ça, c'est le 1er point et pour l'instant on on n'y va pas le 2ème point, moi j'ai j'ai lu l'amendement de Madame Garnier, qui dit : cette mesure n'apparaît pas justifiée au regard des gains extrêmement limité en terme de production d'énergie qu'on peut en attendre, une priorité aux bâtiments de France par rapport à l'enjeu patrimonial, puisqu'on est sur des injonctions contradictoires puisque toute manière on est sur des productions qui sont pas sur l'équilibre du réseau électrique français expliquez moi : dans ce cas-là, l'avis conforme qu'on a voté hier, parce que l'avis conforme qu'on a voté, hier, qui est, je me permets de le dire du strictement grand n'importe quoi, on a donné à des individus, la capacité de décider de la totalité de la stratégie énergétique 2 régions complet puisque ce qui est écrit dans l'amendement et pas dans l'objet, c'est 10 kilomètres autour du bâtiment historique en Bretagne,

d'éolien, donc ça n'est pas possible de donner à quelques individus, le droit de décider la stratégie énergétique d'une région entière, alors que l'État dit aux régions dans le même temps, vous devrez tenir des objectifs quantitatifs, donc je trouve que, l'avis conforme l'avis conforme ici parce que ça ne joue pas sur beaucoup de production électrique entend mais on a voté strictement l'inverse hier. Pardon, mon cher collègue, mais il y a, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre traiter des agents de l'État d'individus comme si prenait des décisions seul, vous savez, mon cher collègue qui a une historique de la législation du Patrimoine en France, c'est une fierté que nous avons, d'avoir construit au fil du temps, des dispositifs de protection de notre Patrimoine, et c'est bien ça qu'on saisit les communes, toutes les communes, on voit bien ce que sont en train de faire de nombreuses communes de protéger leur Patrimoine pour mieux mettre en valeur leur identité et développer leurs capacités aussi touristique, moi je veux bien qu'on qu'on discute entre soi de de tous les avantages de l'énergie renouvelable, je suis favorable à l'énergie renouvelable, mais il faut qu'on soit conscient que l'énergie renouvelable, se heurte à des réactions fortes de nos concitoyens et notamment dès lors qu'il atteint le Patrimoine il y avait une un équilibre qui était, me semble-t-il, dans le texte initial du gouvernement, qui était de dire développons l'énergie renouvelable, mais faisons attention au Patrimoine en ne touchant pas aux mesures de protection, il s'avère que. Il y a eu débat c'est normal je j'ai au niveau de la commission et qu'il y ait eu une un un moment une réflexion sur le rôle des ABF je, je, je, je, je le comprends mais néanmoins, je crois qu'il faut revenir à l'équilibre de départ qui est de dire ne toucheront pas aux dispositifs de protection existantes, c'est tout le sens de des 2 amendements que évidemment je je je je soutiens entièrement je crois que ce que nous a dit la ministre sur la la l'instruction qui est en cours d'harmoniser les les points de vue était une dimension extrêmement importante, je crois qu'il ne faut pas tomber dans dans ces excès dans des dans des débats, c'est pas le le le l'intérêt du rôle de la BF la ABF joue un rôle fondamental dans la protection du Patrimoine, c'est le fait que d'un département à l'autre, on ne comprennent pas forcément c'est ça la question que vous posez, mes chers collègues, passer d'un avis conforme à un avis simple ça ne répond pas à cette question, la la réponse à cette question, c'est l'instruction sur lequel les services de l'État sont en train de travailler sur lequel évidemment nous au niveau de la commission culture, nous serons très attentifs et donc j'invite vraiment chacun à soutenir les les 2 amendements de suppression. Monsieur Gremillet. Oui, merci Monsieur le Président, c'est, c'est effectivement un sujet. Et je remercie notre collègue. Et je partage, je suis un peu rassuré d'entendre qu'effectivement on est proche d'un cadre de règles de mais surtout d'un cadre national concernant cette richesse du Patrimoine sur nos territoires. Mais il y a un autre point que je voudrais poser. Je suis pas sûr que ça soit incompatible. Cette protection. Avec aussi un enjeu tout ce qui est renouvelable n'est pas forcément incompatibles systématiquement avec la protection je dis ça parce que il il faut dépassionner un peu on on peut, on n'est pas à part, on est dans une société qui évolue et ce Patrimoine cette richesse patrimoniale et elle évolue aussi dans ce contexte là. De nos territoires. Bien sûr, ça remet pas en cause l'amendement qui est proposé, mais ce débat que nous avons à cet instant, je trouve et apaiser en plus je trouve non mais sincèrement, quand vous êtes sur le terrain, on est tous sur le terrain. on a tous des cas. D'où l'importance d'avoir ses règles et le sujet que nous évoquons, là il doit pas le mettre il doit pas être mis en opposition avec la protection du Patrimoine et la vie de la BF, c'est pour ça que je j'insiste le renouvelable, il peut parfois très bien se conjuguer avec il y a peut-être une réflexion à poursuivent là-dessus. Merci monsieur le président, je voulais vous dire moi j'étais partagé au départ sur les amendements qui nous sont proposés, parce que c'est vrai qu'on a tous eu dans nos départements, des difficultés parfois à faire évoluer le sujet et puis je me suis remis dans le dossier, moi je suis sénatrice de la Vendée, et j'habite aux sables d'Olonne et à une époque, hé bien le Patrimoine a été vraiment saccagé pour faire du logement, donc aujourd'hui, je suis persuadé qu'on peut faire de des énergies renouvelables avec le Patrimoine, il faut absolument qu'on arrête d'opposer les choses, comme le disait notre collègue Gremillet, donc l'année l'équipe, la question n'est pas tant avis conforme ou à vie simple la question, c'est comment on va réussir à gérer dans les départements, non pas l'ABF, mais toutes ces ABF qui se prononce à géométrie variable et qui parfois retard oui il faut le dire retarder des projets donc si notre collègue Françoise Gatel était là, il a été question tout à l'heure avec Rémy Pointereau, des petites cités de caractère, on ne peut pas imaginer aujourd'hui saccagée aussi peut être à cause d'un avis simple les petites cités de caractère qui sont dans nos territoires, des outils de dynamisme économique, de revitalisation des centres-villes et des centres bourgs, donc pour toutes ces raisons, hé bien mon cheminement fait que je vais bien entendu voter les amendements qui nous sont proposées, je vous remercie. en tant que mère et j'ai une fois déposé un permis de construire auprès de la BF pour transformer une ancienne fermette logement social 1er permis retoqué la BF nous donne ses prescriptions, 2 mois après, je reviens avec la deuxième permis avec prescription refusé, elle me rend sa nouvelles prescriptions je reviens avec le 3ème, identique au 1er permis et là le valide à un moment donné à moi que je l'ai peut-être usé quand même poser des questions sur la la réflexion que parfois les ABF peut avoir 2ème réflexion hier soir suite à l'attention de mon collègue de la Somme, j'ai évoqué, moi le, le Patrimoine mondial classé le bassin minier Nord-Pas-de-Calais Patrimoine mondial classé à l'UNESCO et moi je suis maire d'une commune, parce que c'est le Nord et Pas-de-Calais, donc moi la commune dans le Pas-de-Calais, j'ai une cité minière, c'est la même rue, je traverse la rue, je change de trottoir je change de communes, mais en plus je change de département, donc à un moment donné, comment voulez-vous avoir un avis de la BF pour la rénovation de ces logements en fonction des couleurs puisque l'ABF du Pas-de-Calais n'est pas en accord avec la bf du Nord, donc à un moment donné, comme l'a dit Madame, une milice vivement qu'il y ait une charte niveau national puisque, entre les départements, les Abesses puissent accorder leurs violons. Monsieur Folliot. Merci monsieur le président, mes chers collègues, la France, c'est la première destination touristique au niveau mondial et comme cela a été dit par un certain nombre de nos collègues, ceci est somme toute la résultante de ce qui a été fait par nos anciennes depuis des décennies et et nous avons tous en mémoire la loi Malraux qui a changé beaucoup de choses pour notre pays et qui a été un élément fondateur parce qu'il y a eu cette prise de conscience de la nécessité de préserver ce Patrimoine moi je rejoins ce que dit tout à l'heure notre collègue Pierre Ouzoulias et et et ce qu'on dit aussi nombre de nos collègues, c'est un enjeu essentiel et fondamental et que dans ce cadre-là, il est important et essentiel que nous puissions nous projeter avec cette même vision, on le voit d'autres pays n'ont rien fait, ils ont totalement saccagé tout leur Patrimoine, on pense à la Chine et il y a quelques autres pays parce que il n'y avait pas ces outils juridiques de protection du Patrimoine et donc je crois que c'est un élément essentiel, si je prends un exemple dans mon département, la cité épiscopale d'Albi n'aurait jamais été classée au Patrimoine mondial de l'humanité, si nous n'avions pas pris à l'époque un certain nombre de dispositions législatives pour protéger alors parfois de manière un peu stricte, c'est vrai et il y a des propos qui ont été tenus par les uns et par les autres au regard de décisions d'architecte des Bâtiments de France, que nous avons peut-être subi dans nos vies communal et pour lesquels nous n'avons pas toujours compris, faisons leur confiance, ils sont dépositaires, je veux dire à certains égards de de certains éléments collectif et et donc de cet objectif de, préservation du Patrimoine, qui est un élément est essentiel et fondamental, alors c'est vrai qu'il y a des situations qui sont différentes, on ne pourra pas harmoniser au niveau national pour une bonne et simple raison, c'est que la situation est très différente d'une commune à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre et donc faisons-leur confiance confiance par rapport à ça parce que je ne crois pas qu'il y est, le schéma d'abus de pouvoir de l'architecte des Bâtiments de France, il y a simplement une volonté de leur part d'essayer de s'inscrire positivement dans une démarche qui est une démarche collective est fondamentale, essentielle qui est celle de la préservation de notre Patrimoine, je vous remercie.

Non, mais je ne veux pas je veux privé la parole à personne Madame Robert. Merci monsieur le président je vais être rapide, mes chers collègues, d'abord je voudrais remercier le rapporteur Mandelli et Madame la Ministre, pour leur avis favorable et si effectivement le travail interministériel qui est en cours et aboutit à une forme en tout cas de charte qui permet d'homogénéiser et d'harmoniser les choses et si ça, ça a permis en tout cas d'emporter l'avis favorable, je m'en réjouis et je vous en remercie, vous dire une chose : j'ai l'impression de revivre les débats de la loi élan j'ai l'impression de revivre les débats chers collègues Pointereau lorsque vous avez déposé votre proposition de loi avec notre collègue à l'époque sur la revitalisation des centre-bourgs sur la question Patrimoine versus finalement autre politique, je crois qu'il faut qu'on arrête parce qu'on a eu tous des expériences malheureuses du rouleau douloureuse avec nos ABF mais arrêtons de faire des cas particuliers,

d'abord c'est un corps d'état qui travaille avec le ministère de tutelle qui ne forcément qui qui est là aussi et on l'a vu sur la question du Patrimoine pour mettre des garde-fous pour discuter avec les élus, vous savez, moi j'aurais bien voulu qu'on ait les mêmes garde-fou pour les entrées de ville parce que à un moment donné il y a aussi des élus qui pourraient penser aussi différemment les entrées de ville et souvenez-vous de cette de de cet article, la France moche, oui, il y a vraiment un un travail à faire sur les entrées de ville et on, on le sait très bien, donc il faut qu'on arrête ces débats et j'ai, je sais que depuis la loi élan parce qu'on a ouvert une brèche parce qu'on a ouvert une brèche sur la question des des ABF, hé bien on va de nouveau sûrement dans les années qui viennent à avoir de nouveau ces ces débats avec les ABF mais arrêtons vraiment et et au contraire, on peut se féliciter d'avoir ces personnes qui, à un moment, Me ces garde-fou, mettez l'eau on peut les mettre autour de la table sans considérer qu'obligatoirement ce ce soit un véto c'est un avis conforme effectivement mais un moment donné, ce sont des personnes qui ont dans l'échange avec les élus ou les porteurs de projets peuvent aussi convenir qu'à un moment, c'est possible, et donc ne vont pas mettre en place leur avis conforme, je trouve que vraiment on est dans un chômage arrête mais vraiment votons mais je m'en félicite. Madame Préville. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons un devoir de préservation du Patrimoine, dont nous avons hérité, et ceci pour ceux qui après nous viendrons c'est notre responsabilité, je vous parle d'un département, le Lot, dont l'attractivité est principalement due à son Patrimoine je vous citerai la ville de Figeac et le village de Rocamadour, la première destination touristique mondiale et donc un enjeu économique important pour la France et qui sommes-nous finalement dans notre histoire, vieille de 2 1000 ans pour en quelque sorte tout sacrifier au prétexte de notre consommation des d'électricité, la situation est complètement nouvelle, parce que nous allons avoir effectivement beaucoup d'installation, c'est le principe de ces énergies renouvelables, qui ne produisent pas en quantité et que donc nous avons un devoir très important de préservation nous humanité nous avons besoin aussi de ces endroits préservés, qui sont exempts de cette modernité et préserver ses espaces de beauté, qui sont des îlots intemporel contre ses installations qui vont se faire partout pour nos enfants, nous devons laisser l'expérience que nous avons une ou deux ces espaces que nous avons pu connaître préserver je vous remercie. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, je crois qu'ici tous dans cette assemblée, nous sommes très attachés à notre Patrimoine, bien entendu, et nous en tant qu'écologiste, lorsque nous avons essayé de faire sortir un peu les villes des coeurs, les voitures, excusez-moi, les voitures des coeurs des centre-ville effectivement c'est aussi une préservation du du Patrimoine, mais on a sans doute des visions un peu différent un peu différent du Patrimoine il y a le Patrimoine vivant il y a le poitrine moines qui peut être fossilisé musée y fiez il faut faire attention à tout cela il y a des gens qui vivent au autour des bâtiments historiques, ces gens-là effectivement sont dans la société et donc. peuvent être en attente aussi d'évolution et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à de tels défis de tels, de tels enjeux, que, hé bien il faut que nous avancions de concert et j'ai bien entendu la ministre qui disait tout à l'heure qu'il a, il y a la charte qui est en cours mais dans combien de temps va-t-elle aboutir donc pendant ce temps là, hé bien nous allons confier le développement des énergies renouvelables à quelques personnes qui font sans doute très bien leur travail, mais qui le font avec une focale qui est à mon avis, parfois un peu étroite, donc il faut absolument aller pour l'instant et je continue de défendre vers un avis simple parce que cet avis conforme donne trop de pouvoirs avec une focale restrictif, combien de fenêtre de toit, combien d'isolation par l'extérieur, combien de doubles vitrages ont été interdits pendant des années, qui ne préserve pas l'avenir et qui surtout sont inconfortables pour de nombreux habitants, je pense qu'il faut prendre tout ça en compte, il y a des gens qui vivent autour des bâtiments historiques et il y a une société autour des bâtiments historiques.

opposer d'une certaine façon, préservation du Patrimoine et préservation de l'environnement, or, or le Patrimoine fait partie de l'environnement, il est partie prenante de l'environnement, voilà donc on doit pouvoir se retrouver avec un petit peu d'ouverture d'esprit. Que marchand et ensuite on passera au vote sur la. évidemment. Très rapidement, je pense que s'il fallait conclure notre débat moi je j'en appellerai à Jaurès, faut aller vers l'idéal, mais il faut comprendre le réel et comprendre le réel, c'est à voir effectivement perspective que la préservation de notre Patrimoine, c'est l'affaire de tout le monde c'est l'affaire effectivement de de tous les élus locaux que nous avons été et moi je donne crédit effectivement aux propos de Madame le ministre et aux propos du rapporteur sur cette mission conjointe qui est menée pour faire en sorte bien les points de vue des uns et des autres puissent se rejoindre pour faire en sorte que nous allions ses 2 priorités que sont à la fois, énergies renouvelables et préservation de notre Patrimoine. Bien, on va passer au vote juste en disant que monsieur Jaurès n'a jamais opposé le réel à l'idéal il il y avait pas de mais chez Jaurès entre l'idéal et le réel mais enfin. Commentaires personnels or compte rendu parce que le président n'a pas le droit d'en faire donc nous allons voter sur. Sur les deux amendements donc qui et pour les 2 amendements. Qui est contre.